La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 février 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue, Jean-François Voguet, qui fut sénateur du Val-de-Marne de 2004 à 2011. de 2004 à 2011. Le débat à la suite du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes aura lieu le mercredi 24 mars 2021, à seize heures quarante-cinq. Dans l'organisation de ce débat, nous pourrions attribuer, après la présentation du rapport par le Premier président de la Cour et les interventions des commissions des finances et des affaires sociales, un temps de parole d'une heure pour les groupes politiques. En conséquence, le débat préalable au Conseil européen, initialement prévu le mercredi 24 mars 2021, serait avancé au mardi 23 mars 2021, le soir. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote, en deuxième lecture, sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine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

la singularité de la France s'exprime au travers de la richesse et la diversité de son patrimoine. Il touche à ce que nous sommes. Il est une part de notre identité, de notre mémoire et, donc, de notre culture commune. Au-delà, c'est un fort levier de croissance et d'emplois. Il contribue ainsi à l'attractivité de nos territoires. Je sais que le Sénat est très attaché à ce patrimoine. Il nous incombe collectivement de le protéger, de le valoriser et de le restaurer.

Depuis sa création, le ministère de la culture contribue à cette préservation du patrimoine. Il n'est pas seul dans cette action, car il a pu compter, au fil des années, sur des partenaires essentiels. Je pense bien sûr aux collectivités territoriales, mais également aux fondations, parmi lesquelles la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine a su développer son action en engageant des campagnes de souscription publique, de financement participatif, en mobilisant le mécénat d'entreprise ou en délivrant son propre label. Dès sa création, l'État lui a en effet confié la mission de délivrer un label en faveur du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, label qui donne droit à un régime de déductions fiscales au titre de l'impôt sur le revenu. La Fondation a aussi contribué à l'initiative du loto du patrimoine, souhaité par le Président de la République, dont le succès ne se dément pas et dont elle continue à assurer le pilotage, en lien avec la mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern et les directions régionales des affaires culturelles.

promulguée en juillet dernier, a repris la disposition que vous proposiez. Cela a permis une accélération de sa mise en oeuvre, ce dont nous pouvons collectivement nous réjouir, mais a rendu, de fait, l'article 1 sans objet.

sur la possibilité pour la Fondation de réaffecter des dons devenus sans objet en raison de la caducité des projets ou de leur financement en intégralité, la Fondation a su trouver une solution. L'article reste donc supprimé.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme d'une lecture dans chaque assemblée, le parcours législatif de la proposition de loi déposée par notre collègue Dominique Vérien, voilà bientôt deux ans, pour améliorer l'efficacité de de la Fondation du patrimoine est presque achevé. Je dis « presque », car il faudra une ultime lecture à l'Assemblée nationale pour valider les deux coordinations que nous avons adoptées en commission il y a treize jours. La commission a en effet estimé que, sur le fond, le texte que nous avait transmis l'Assemblée nationale à l'issue de ses travaux en première lecture constituait un excellent compromis. nationale a souscrit à l'essentiel des dispositions du texte, n'y apportant, au final, que très peu de modifications substantielles. Elle a totalement adhéré aux principales orientations que nous avions eu à coeur de défendre en première lecture, notamment celle de faire en sorte que cette réforme ne détourne pas la Fondation du patrimoine de son coeur de métier : le soutien à la protection du patrimoine rural. L'Assemblée nationale a dit « oui » à l'assouplissement des conditions de délivrance du label de la Fondation ; « oui » à l'éligibilité des parcs et jardins à l'extension de son périmètre géographique aux sites patrimoniaux remarquables, aux sites classés au titre du code de l'environnement et à toutes les communes de moins de 20 000 habitants. Elle a même complété notre dispositif sur deux points : d'une part, elle a précisé que seule la labellisation des immeubles non habitables « caractéristiques du patrimoine rural » échappait à toute condition de périmètre géographique d'autre part, elle a souhaité autoriser les propriétaires dont le bien ne serait pas visible de la voie publique, mais qui s'engageraient à le rendre accessible au public, à bénéficier des mêmes avantages fiscaux. L'Assemblée nationale a également validé la réforme du conseil d'administration, qui permet de réduire le nombre de ses membres afin de le rendre plus opérationnel et de rapprocher sa composition de celle du droit commun des fondations reconnues d'utilité publique, malgré une différence notable : le maintien de la moitié des sièges aux représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs, afin de préserver leur confiance dans le fonctionnement de la Fondation et de les inciter à la soutenir davantage. L'Assemblée nationale n'a pas non plus vu d'obstacle à la suppression des prérogatives de puissance publique dont disposait la Fondation, et dont elle n'a jamais fait usage. La seule légère déception suscitée par le texte transmis par l'Assemblée nationale, c'est peut-être la suppression de l'article 5, qui mettait en place un mécanisme à portée rétroactive facilitant la réaffectation, par la Fondation, à un autre projet, des dons devenus sans objet, soit parce que le projet pour lequel ils avaient été collectés serait devenu caduc, soit parce qu'il aurait déjà été intégralement financé. Le but de cette disposition était de permettre à la Fondation de réaffecter plus facilement les 10 millions d'euros qui sont aujourd'hui immobilisés dans ses caisses, faute d'être parvenue à obtenir l'accord des porteurs de projet initiaux pour leur réaffectation. Les fragilités juridiques de ce dispositif, que nous avions nous-mêmes identifiées en première lecture, ont conduit l'Assemblée nationale à préférer l'abandonner, aucune rédaction alternative ne s'étant révélée possible. La commission de la culture s'est ralliée à cette suppression, dans la mesure où la Fondation du patrimoine nous a indiqué qu'elle avait bon espoir que la situation se règle à plus ou moins long terme, même en l'absence de disposition juridique. L'un de ses bénévoles s'est en effet porté volontaire pour contacter tous les porteurs de projet dont les dons doivent être réaffectés. Il s'agira bien sûr d'une entreprise de longue haleine, mais nous nous emploierons à surveiller de près l'évolution de la situation dans les années à venir. Malgré cet accord global sur le fond du texte, la commission a été contrainte d'adopter deux amendements de coordination. amendement concerne l'article 1, dont les dispositions ont été intégrées à l'identique dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020, en juillet dernier. L'objectif était de permettre une entrée en vigueur plus rapide de la réforme du label afin de contribuer à la relance de l'activité du secteur des patrimoines.

La seconde coordination que nous avons effectuée concerne l'article 1 , inséré par les députés pour remplacer dans l'un des articles du chapitre du code du patrimoine consacré à la Fondation une terminologie obsolète faisant référence aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une appellation qui n'est plus utilisée depuis 2005. Ils avaient malencontreusement omis d'effectuer le même remplacement un peu plus bas dans l'article. Nous en avons profité pour nettoyer toutes les références à l'inventaire supplémentaire qui subsistaient dans les parties législatives des codes. Tous les autres articles ont fait l'objet d'adoptions ou de suppressions conformes. Ces coordinations rallongent malheureusement le temps de la navette parlementaire, mais il n'était pas possible de nous y soustraire. Il nous reste à souhaiter que l'Assemblée nationale trouve un créneau dans son ordre du jour d'ici à l'été, car ce texte, même amputé de son article phare, déjà entré en vigueur, conserve des dispositions essentielles pour permettre à la Fondation de mieux se projeter vers l'avenir et d'avoir une action toujours plus efficace en faveur de la protection du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques. La parole

aux côtés des grands monuments historiques que nous connaissons tous se tient une myriade de monuments plus discrets : moulins, fontaines, anciennes manufactures, chapelles, colombiers, bateaux de pêcheurs, lavoirs Ce petit patrimoine de proximité fait le charme de nos villes et de nos villages, mais il connaît aussi les affres du temps et nécessite régulièrement des actions de sauvegarde et de restauration. La Fondation du patrimoine est ce grand hôpital dans lequel des milliers de projets locaux de sauvegarde voient le jour. La Fondation agit au plus près des besoins, avec un réseau de 22 délégations régionales et de 100 délégations départementales, animées par 600 bénévoles présents sur le terrain. Nous avons vu sa puissance après le désastre de l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. En quelques jours, la Fondation du patrimoine a levé l'équivalent d'une année de dons. Son action ne s'arrête pas là, tant s'en faut. En 2019, elle a mobilisé la générosité de 280 000 donateurs et de 6 000 entreprises mécènes. favorise l'accès à la culture au plus près de chez soi et renforce le lien intergénérationnel : restaurer et conserver notre patrimoine local, c'est permettre la transmission d'une histoire et d'une identité à nos enfants et petits-enfants. au développement de l'économie et à l'insertion sociale de personnes éloignées de l'emploi, grâce aux nombreux chantiers de restauration. Ses moyens d'action sont de trois ordres la labellisation de travaux ouvrant droit à un avantage fiscal et à un ensemble d'aides ; les campagnes de souscription publique et le mécénat d'entreprise. La proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture au Sénat vise à améliorer l'efficacité de la Fondation du patrimoine, créée en 1996 sur une initiative sénatoriale. Il s'agit, d'une part, d'en rénover la gouvernance, jugée pléthorique, et, d'autre part, d'actualiser les conditions de délivrance du label. Je salue cette proposition de la sénatrice Dominique Vérien. En tant qu'élu d'un département rural, je mesure particulièrement l'importance du soutien de la Fondation du patrimoine aux initiatives locales de restauration du patrimoine de proximité, que nous pouvions autrefois soutenir directement en mobilisant la réserve parlementaire. L'article 1 étendait le périmètre de la labellisation au patrimoine situé dans des communes de moins de 20 000 habitants, contre 2 000 actuellement. Cette disposition, adoptée entre-temps dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative, a été supprimée. En première lecture, le Sénat a adopté une mesure importante prévoyant que la moitié au moins des labels attribués par la Fondation doive concerner des projets de restauration d'immeubles appartenant au patrimoine rural. L'Assemblée nationale a, de son côté, assoupli les conditions d'octroi du label en précisant que les propriétaires s'engageant à rendre leur bien accessible au public pourraient en bénéficier au même titre que les propriétaires dont le bien est visible depuis la voie publique. L'article 3 réforme la composition du conseil d'administration de la Fondation en resserrant le nombre de ses membres et en associant plus étroitement les mécènes et les communes rurales. Il était également proposé à l'article 5 un mécanisme de réaffectation des dons non utilisés. Je regrette sa suppression, bien que je comprenne les risques d'inconstitutionnalité qu'il présente. La Fondation du patrimoine possède l'équivalent de 10 millions d'euros immobilisés à cause de l'abandon de projets. Ces fonds pourraient bénéficier à d'autres projets, mais, en l'absence d'un tel mécanisme de réaffectation des dons, il faudra déployer des moyens importants pour contacter les porteurs de projet afin de recueillir leur accord sur la réaffectation des sommes versées. Cette proposition de loi permettra à de nombreux projets de restauration du petit patrimoine rural de voir le jour. Le label ainsi modernisé contribuera à sauver de la ruine et de l'oubli des édifices emblématiques, tels que certaines églises rurales, joyaux de l'art gothique retraçant des siècles de savoir-faire, dont nous avons la responsabilité. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte vise à faciliter la gestion de la Fondation du patrimoine, à lui redonner du souffle, mais aussi à apporter de la pertinence au label. Le groupe écologiste accueille favorablement la réforme de son conseil d'administration, qui permettra, d'une part, de donner une meilleure place aux structures engagées et actives dans la Fondation et, d'autre part, d'atteindre plus facilement le quorum pour remplir plus efficacement ses missions. Je souhaite saluer également une mesure prévue à l'article 1, finalement intégrée à la dernière loi de finances rectificative, qui redonne à la Fondation un périmètre d'action correspondant au sens de sa mission. Elle pourra dorénavant intervenir sur l'ensemble des communes de moins de 20 000 habitants. Ce périmètre avait été restreint, à l'excès, par une instruction fiscale ; il sera dorénavant bien plus cohérent avec les objectifs de la Fondation. regrettable qu'aucune solution législative n'ait pu être trouvée pour permettre de réaffecter les fonds bloqués de la Fondation, qui représentent tout de même 10 millions d'euros. Cette proposition de loi aura permis de mettre en lumière ce problème, mais d'autres leviers devront être actionnés rapidement pour le régler. Je me permets également de souligner un point de vigilance.

Ces pouvoirs étaient, certes, inhabituels pour une structure de ce type, et ils n'avaient jamais été mis en oeuvre. Mais était-ce une raison suffisante pour lui retirer toute possibilité de les utiliser dans le futur ? Au moment de sa création, il était envisagé que la Fondation du patrimoine puisse jouer un rôle dans l'acquisition, la gestion et la protection de sites naturels, actions pour lesquelles ces pouvoirs exceptionnels auraient pu être utiles et justifiés. L'action de la Fondation est aujourd'hui très peu tournée vers le patrimoine naturel, qui est pourtant particulièrement menacé et qui manque de financements. La protection des paysages et sites naturels remarquables a toute sa place dans la politique du patrimoine. Je regrette donc que cette dimension de son action ne soit pas remise à l'ordre du jour. Toutefois, le groupe écologiste votera cette proposition de loi en raison des avancées positives et concrètes qu'elle apporte.

Madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice Vérien, autrice de la proposition de loi, mes chers collègues,

Cette structure essentielle vient aider financièrement les propriétaires, qu'il s'agisse de collectivités, de particuliers ou d'associations, qui s'investissent pour préserver notre patrimoine de proximité non proximité non protégé, celui de nos centres-bourgs et de nos centres-villes. Élue de la commune de Saint-Pabu, dans le Finistère, je conclurai d'ailleurs en évoquant un exemple concret à quelques pas de chez moi. Par quels moyens cet accompagnement se fait-il ? Par des dons, du mécénat, des aides fiscales, des subventions de collectivités, des jeux, aussi, notamment grâce à la mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern et la Française des jeux, et, enfin, par des apports de la Fondation du patrimoine elle-même. Au total, ce sont près de 3 000 projets par an qui sont portés par cette institution. La proposition de loi déposée par notre collègue du groupe Union Centriste, Mme Dominique Vérien, porte sur la modernisation de la gouvernance et des outils de collecte de cette personne morale de droit privé, reconnue d'utilité publique. un texte bienvenu, que nous soutenons avec mon groupe, et qui va bientôt être définitivement adopté après accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Que notre collègue en soit félicitée L'objectif est, tout d'abord, de rendre plus efficaces les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation confiées à la Fondation du patrimoine. Toutes et tous ici, nous connaissons l'attachement de nos concitoyens à cette identité territoriale, à la nécessité de l'entretenir et, en même temps, les difficultés que rencontrent celles et ceux, notamment les élus locaux, qui sont impliqués dans ces entreprises de conservation.

Parmi les outils à la disposition de la Fondation, que j'évoquais en introduction, il y a le lancement des souscriptions populaires. Les porteurs de projet peuvent en effet solliciter la Fondation pour recueillir des dons, ce qui donne lieu à défiscalisation, mais certains projets n'aboutissent pas ou, alors, ils aboutissent avec d'autres sources de financement. La conséquence, c'est que l'argent ainsi collecté n'est pas dépensé. De façon opportune, la proposition prévoit un mécanisme pour débloquer ces sommes- 10 millions d'euros sont éligibles -, afin de les réaffecter à d'autres projets patrimoniaux. Ces mesures vont bien dans le sens d'une meilleure protection et de la valorisation du patrimoine de proximité. En conclusion, j'aimerais revenir quelques secondes dans le Finistère pour évoquer la restauration et la sauvegarde de l'église Saint-Tugdual, dans la commune de Saint-Pabu, commune où je suis élue depuis de nombreuses années.

du projet, lequel a connu des transformations. Ainsi, au second semestre de 2022, avec l'action de la Fondation du patrimoine, une nouvelle étape de restauration sera entreprise. À quelques kilomètres de chez moi se dresse un autre trésor : le phare de l'île Vierge, plus haut phare d'Europe, plus haut phare du monde en pierre de taille et quatrième plus haut phare du monde,

qui va du château au petit pigeonnier rural, en passant par ses jardins remarquables. Nous savons combien la préservation et la valorisation de ces biens sont essentielles à l'attractivité de nos territoires. Une grande partie de ce patrimoine échappe cependant à la politique de restauration menée au titre des monuments historiques. Aussi, la Fondation du patrimoine est devenue, depuis sa création en 1996, un partenaire privilégié et complémentaire des politiques de protection patrimoniale de l'État.

En effet, chaque année, la Fondation s'emploie à sauver plus de 2 000 monuments non protégés- églises, théâtres, moulins, musées, et même des phares, comme nous venons de l'entendre -, participant ainsi activement au développement économique des centres-bourgs, à la transmission des savoir-faire artisanaux et à l'essor du tourisme rural. J'en profite pour saluer le travail de tous les acteurs, notamment des quelque 600 bénévoles, qui s'investissent dans nos régions, dans nos communes, pour sélectionner les chantiers et mobiliser les financements. Ils font bien souvent dans la dentelle, une approche qui légitime la Fondation, dont je rappelle le statut d'utilité publique. Pour autant, la Fondation doit garder un cap : il s'agit de s'intéresser en priorité au patrimoine non protégé, en particulier au patrimoine rural. Dans cette perspective, la proposition de loi offre de nouvelles garanties pour renforcer les actions de mise en valeur du patrimoine local. Parmi celles-ci, on ne peut qu'adhérer à la réforme du label « Fondation du patrimoine », qui donne droit à un avantage fiscal incitatif pour la restauration du patrimoine, dont une instruction administrative de 2005 était venue limiter la portée en le réservant au patrimoine rural des villes de moins de 2 000 habitants. Aussi, notre groupe est favorable à l'élargissement du bénéfice potentiel du label à tous les immeubles situés dans des communes de moins de 20 000 habitants, un seuil qui correspond mieux aux nouveaux contours du monde rural.

le savoir-faire français en matière d'aménagement paysager étant également un élément très reconnu et apprécié de notre patrimoine culturel. Je tiens à rappeler le travail d'amélioration de ce texte effectué par le Sénat lors de sa première lecture. Ainsi, l'objectif de sauvegarde du bâti rural a été renforcé

nos collègues avaient élargi le collège des collectivités territoriales aux communes rurales. Tout cela va naturellement dans le bon sens ; notre groupe y souscrit pleinement. S'agissant de la gouvernance de la Fondation, les orateurs précédents ont déjà rappelé que le texte vise à la moderniser, à la simplifier et à la rendre plus efficace pour la rapprocher du droit commun des fondations reconnues d'utilité publique. Plus précisément, la rédaction proposée par le Sénat devrait permettre de fluidifier les décisions, objectif que je partage évidemment. Le seul regret que je souhaite évoquer concerne la question des ressources financières mises à disposition de la Fondation. L'article 5, qui offrait dans le texte initial la possibilité de réaffecter des dons à un autre projet en cas de non-réalisation des travaux financés, a été supprimé par l'Assemblée nationale ; nos collègues députés ont mis en avant la fragilité juridique du dispositif. argument, mais le retrait de cet article ne doit pas empêcher le Gouvernement de réfléchir à une base légale qui permettrait d'éviter le blocage de fonds. Doit-on s'inquiéter aussi, dans le contexte économique actuel, d'une possible raréfaction du mécénat des entreprises, vecteur sur lequel s'appuie la Fondation ? Peut-être, madame la ministre, disposez-vous d'éléments sur ce risque ? Mes chers collègues, ici, dans la maison des collectivités locales, il n'est pas besoin d'en dire davantage pour convaincre de la nécessité de sauver le petit patrimoine du quotidien, d'entretenir les bâtis caractéristiques de nos campagnes, qui irriguent la vie locale et font le charme des détours sur les routes de France. Le RDSE, comme je l'ai expliqué, est favorable aux aménagements proposés autour de la Fondation du patrimoine. Par conséquent, nous voterons ce texte avec enthousiasme.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la Fondation du patrimoine a été conçue en juillet 1996 la volonté politique assumée de créer un outil expérimental qui puisse suppléer l'action publique par le recours à la mobilisation de l'activité de bénévoles, au mécénat d'entreprise et à la générosité privée. demeure aujourd'hui un hapax : c'est le seul organisme privé indépendant à but non lucratif dont le statut est fixé par la loi et dont le financement repose, en grande partie, sur une recette domaniale de l'État qui n'est pas soumise au contrôle budgétaire du Parlement. À la fin du précédent millénaire, dans l'euphorie des réflexions alors menées sur la réforme de l'État, la Fondation du patrimoine devait être le laboratoire de la collaboration heureuse entre partenaires publics et privés et constituer ainsi un utile auxiliaire de l'État dans son action en faveur du patrimoine rural non protégé.

ans plus tard, ce dessein novateur a été oublié et ce projet ambitieux apparaît comme une chimère. La Fondation du patrimoine ne compte que 6 000 adhérents et dispose d'un budget de 32 millions d'euros. Ses membres espérés et jamais venus ont finalement été remplacés, plus adéquatement, par les acheteurs d'un billet du loto du patrimoine. Comme le souligne la Cour des comptes, la Fondation du patrimoine n'a jamais encouragé l'adhésion directe des personnes physiques, estimant qu'elle n'aurait pas les moyens d'assurer l'organisation et la promotion du réseau qu'elle aurait pu constituer. Par ailleurs, dépourvue des ressources privées qu'elle espérait, la Fondation du patrimoine a finalement été sauvée, en 2003, par l'affectation d'une fraction du produit des successions appréhendées par l'État pour cause de déshérence. Cette ressource erratique représentait, en 2010, 40 % de ses revenus. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2013, souligne justement que cette recette domaniale de l'État échappe au contrôle du Parlement, en contradiction avec l'article 51-1 de la loi organique relative aux lois de finances, qui fait obligation au Gouvernement d'informer le Parlement des recettes publiques affectées à des personnes morales autres que l'État. À tout le moins, madame la ministre, il serait légitime que le Gouvernement satisfît à cette obligation législative à l'occasion de la prochaine discussion budgétaire. Cet apport d'argent public a certes permis à la Fondation du patrimoine de développer les actions qui étaient sa raison d'être, mais il a eu pour autre conséquence de complexifier ses rapports avec l'État, qui lui a demandé en échange de prendre à sa charge des politiques publiques qu'il ne pouvait plus financer ou organiser. L'ambiguïté de cette relation a été révélée au public lorsque la Fondation a décidé de suspendre sa collecte de fonds en faveur du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame Votre prédécesseur, madame la ministre, avait alors fait part à notre commission de sa perplexité devant cette décision. Elle était pourtant parfaitement légitime, venant d'un organisme dont l'indépendance a été voulue par sa loi fondatrice, mais n'en posait pas moins la difficile question de la relation entre l'État et la Fondation. La présente proposition de loi porte modification du gouvernement de la Fondation du patrimoine et prend ainsi acte de l'évolution de son fonctionnement par rapport au projet d'origine. La mesure est de bon sens ; on peut néanmoins se demander s'il est pertinent de continuer à fixer dans la loi les statuts d'un organisme dont la pratique s'est sensiblement écartée des missions qui lui avaient été assignées en 1996. Dans son rapport d'information du 25 juillet 2002, notre ancien collègue sénateur Yann Gaillard estimait que la Fondation du patrimoine devait « avoir un rôle pilote dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dit " non protégé " C'est pourquoi il avait souhaité, au nom de la commission des finances, la doter de ressources budgétaires pérennes. La Fondation du patrimoine a parfaitement accompli cette nouvelle mission, à proportion des moyens mis à sa disposition. Toutefois, cette évolution aurait dû être accompagnée d'une réflexion d'ensemble sur les objectifs et les moyens d'une politique nationale en faveur du patrimoine rural non protégé. Déjà, en 1987, dans le cadre de la mission Patrimoine 2000, Serge Antoine soulignait que le patrimoine rural avait été l'oublié d'une société ingrate à l'égard de ses agriculteurs.

Je l'avais déjà souligné lors de la première lecture de ce texte, mais je tiens à le faire une nouvelle fois : il ne serait pas ce qu'il est sans le regard compétent, les remarques et les modifications avisées de son premier rapporteur, Jean-Pierre Leleux.

Mais il reste encore la modification du conseil d'administration de la Fondation. Cela pourrait être anecdotique, mais la gouvernance d'une fondation est une chose importante. La Fondation du patrimoine prend de l'ampleur et intervient dans de nombreuses missions, comme le loto du patrimoine. Elle a su prendre tout de suite sa part dans la sauvegarde de Notre-Dame, même si elle a arrêté sa souscription un peu plus tôt que ne l'espérait M. Riester. Enfin, elle est en train de renouveler et de développer le nombre de ses bénévoles dans nos régions. Pour cela, elle souhaite, ce à quoi la Cour des comptes l'y invite avec force, se doter d'une gouvernance plus légère et plus efficace. Je n'ai aucun intérêt personnel dans cette démarche, puisque, à l'issue du parcours de cette proposition de loi, les parlementaires ne siégeront plus

Maintenant, il me reste à vous demander, madame la ministre, de nous aider à aller jusqu'au bout de cette réforme. La Fondation du patrimoine en a besoin, et ce qui est bon pour la Fondation est bon pour le patrimoine ! Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte.

depuis sa création en 1996, la Fondation du patrimoine s'est affirmée comme un acteur incontournable de la préservation d'un patrimoine de proximité, non protégé, mais caractéristique de nos territoires ruraux. La Fondation accompagne chaque année des milliers de projets ; ce sont autant de pépites locales qui participent de l'identité et de l'attractivité des collectivités concernées et doivent être protégées et valorisées Nous connaissons toutes et tous dans nos territoires de tels trésors qui bénéficient de ce précieux appui. Je pense ainsi, pour ma part, au prieuré de Manthes, bâtiment historique remarquable qui est devenu au fil du temps un lieu d'éveil artistique de référence, au pigeonnier qui surplombe le village haut perché de Mirmande, ou encore au salon chinois de l'hôtel Lagier de Vaugelas à Die, lieu trop longtemps oublié : les exemples ne manquent pas à un consensus, en première lecture, autour de la nécessité d'élargir le champ d'action de la Fondation du patrimoine et de moderniser sa gouvernance et sa façon de fonctionner, tout en maintenant son coeur de mission, la sauvegarde de ce patrimoine rural. Je me réjouis que cette vision ait également guidé nos collègues de l'Assemblée nationale. Si, en l'état, la rédaction du texte ne laisse aucune ambiguïté quant au patrimoine ciblé dans ce cadre, l'élargissement du label nécessite, pour être opérant, un effort financier pérenne, point sur lequel nous saurons rester vigilants à l'avenir. La qualité du travail collectif mené autour de l'article 1, mesure phare de ce texte, et la reconnaissance du soutien indispensable que peut apporter la Fondation, aux côtés de l'État et des collectivités territoriales, à la relance de l'activité dans le secteur du patrimoine ont conduit à une adoption anticipée de ses dispositions, dans le cadre de la loi de finances rectificative de juillet 2020. C'est une accélération dont nous pouvons nous féliciter. Ainsi, une fois l'article 1 et l'article 5 supprimés- je reviendrai sur ce dernier dans la suite de mon propos -, la disposition la plus importante introduite par ce texte, à l'article 3, gouvernance de la Fondation et la composition de son conseil d'administration ; elle exprime une volonté de simplification et de gain d'efficacité. Nous avions su trouver lors de nos travaux en commission un point d'équilibre à ce sujet, que je souhaite de nouveau saluer. La composition retenue rapproche la Fondation du statut type des fondations reconnues d'utilité publique ; elle intègre par ailleurs désormais en son sein des représentants des collectivités territoriales et des associations de défense du patrimoine, qui sont des interlocuteurs précieux, car ils agissent au plus près des territoires et des projets concernés. Je conclurai mon propos en revenant sur l'article 5, qui offrait à la Fondation la possibilité de réaffecter des dons versés avant 2015 pour des projets cet article constituait depuis le début du parcours législatif de ce texte un point fort d'incertitude, tant nous craignions que le manque de solidité juridique du dispositif proposé nous expose à une censure du Conseil constitutionnel. Le maintien de la suppression qu'en a faite l'Assemblée nationale s'impose par conséquent comme une décision de sagesse. Il ne nous faut cependant pas oublier les raisons qui ont poussé la Fondation à solliciter en premier lieu un tel outil législatif : l'ampleur de la somme concernée, conjuguée au travail titanesque que représente pour cette structure la quête des anciens donateurs. Si la Fondation du patrimoine a finalement renoncé à une telle disposition, nous devons avoir conscience du coût humain que représente cette recherche : elle requiert une mobilisation bénévole de plusieurs années. Mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de cette proposition de loi, car nous partageons ses objectifs et la vision d'une Fondation du patrimoine résolument engagée en faveur de la préservation et du rayonnement de notre patrimoine rural et et hyper-rural. Espérons que ce riche patrimoine, qu'il nous faut appréhender dans sa dimension aussi bien matérielle qu'immatérielle, pourra continuer à compter sur notre soutien et sur celui du ministère de la culture.

Oui, au Sénat, on aime la Fondation du patrimoine ! On l'aime non seulement parce qu'elle est née d'une initiative sénatoriale, celle d'un de vos compatriotes de Maine-et-Loire, madame la ministre, le sénateur Jean-Paul Hugot,

souvent situé dans les zones rurales. Au Sénat, on salue donc le travail de la Fondation du patrimoine, qui soutient 3 000 projets de sauvegarde publics ou privés, majoritairement dans de petites ou ou très petites communes. Elle peut ainsi se prévaloir d'avoir sauvé, préservé ou protégé quelque 32 000 sites en vingt-cinq ans. À cette fin, elle dispose de plusieurs outils efficaces.

de souscriptions populaires et, plus récemment, du loto du patrimoine, dont elle assure le pilotage et la gestion des recettes. C'est elle, encore, qui a aidé l'État à organiser la souscription nationale pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Enfin, sa capacité d'action est assurée par des bénévoles, qui se chargent de mobiliser le secteur privé et de nouer des partenariats avec les entreprises. La Fondation compte 600 bénévoles. La Cour des comptes, tout en soulignant de la Fondation, a formulé plusieurs recommandations pour développer encore son action. Nous en trouvons la traduction dans la présente proposition de loi, due à l'heureuse initiative de Dominique Vérien, que je tiens à saluer. Comme l'a expliqué notre rapporteur Sabine Drexler, que je remercie pour ses travaux, l'octroi du label de la Fondation sera étendu et facilité. Son périmètre sera désormais inscrit dans la loi, de manière à supprimer les limites fixées

ont le plus grand besoin d'une réhabilitation, ce qui a légitimé un élargissement du label aux communes de moins de 20 000 habitants. Pour autant, le Sénat a garanti que le patrimoine rural demeurerait prioritaire, puisqu'il devra représenter la majorité des immeubles labellisés. Nous avons aussi clarifié le nouveau champ d'application du label, pour qu'il puisse également s'appliquer aux parcs et jardins, aujourd'hui exclus du dispositif. Je tiens à cette occasion à saluer le travail de notre ancien collègue et rapporteur Jean-Pierre Leleux. S'agissant de la gouvernance de la Fondation du patrimoine, il est proposé dans ce texte de réduire l'effectif du conseil d'administration de la Fondation et de rapprocher sa composition de celle d'autres fondations reconnues d'utilité publique. Les travaux du Sénat ont permis de mieux y associer les associations de défense du patrimoine et des représentants des collectivités territoriales, ce qui assurera la représentation des communes rurales et garantira encore une fois le rôle prioritaire de la Fondation dans le soutien au patrimoine de ces petites communes.

notamment pour des équipements culturels au coeur des territoires. Grâce à elle, la friche industrielle est devenue médiathèque ; l'ancienne prison, école de photo ; le mur d'enceinte, chantier d'insertion. Ses missions sont donc culturelles bien sûr, mais également économiques et sociales. En effet, dans cette période de crise sanitaire, les projets de restauration jouent plus que jamais un rôle essentiel de relance économique, en participant au maintien et à la création d'emplois dans les secteurs du bâtiment, des métiers d'art et du tourisme. Nous devons soutenir leur multiplication, au travers de petits chantiers qui permettent de développer la formation et la transmission des savoir-faire de nos artisans et de nos artisans d'art.

! Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. Mes chers

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

et un enjeu financier majeur, à la mesure de la pandémie que nous vivons. Notre débat, mes chers collègues, mérite mieux que des «

! Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit chez les gens de bon sens ... Nous, nous sommes au Parlement, et c'est à nous, avec le Gouvernement, de parler, comme dirait le Premier ministre, « en responsabilité » de ce qui sera fait.

les 70 milliards d'euros de dettes de l'Unédic ne sont pas de même nature que la dette de nos collectivités. La dette de la SNCF, celle qui a été reprise, aussi la nouvelle, celle de 2020, ne sont pas de même nature et n'appellent donc pas les mêmes solutions. Les dettes sous la ligne, principalement les retraites dues

un ménage s'endette en principe pour investir et rembourse ses dettes. Il est surendetté lorsqu'il n'arrive plus à vivre, car ses revenus servent au remboursement de la dette et des charges de la dette.

s'endetter, c'est consommer aujourd'hui le capital de demain. C'est vrai en particulier pour les ressources naturelles. Nous consommons plus vite notre planète lorsque nous nous endettons. Nous faisons payer plus, toujours plus, aux futures générations pour notre propre confort. Avec la dette, c'est le développement durable qui est mis à mal. Je tiens à le dire, parce qu'on

: l'inflation. Est-ce votre solution ? Nous allons en débattre. En tout cas, il y a urgence, car les taux d'intérêt remontent et nous sommes proches de la banqueroute.

Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mesdames, messieurs les sénateurs, nous traversons une crise économique inédite par son ampleur et par sa durée. Pour faire face à cette crise, le Président de la République a fait un choix extrêmement clair : protéger les salariés français et les entreprises françaises, quoi qu'il en coûte. Ce choix s'est effectivement traduit par une augmentation massive de la dépense publique et par un accroissement de notre dette publique, qui atteindra cette année 120 % de notre richesse nationale, contre 98 % en 2019. Ce niveau de dette publique n'avait pas été atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces 20 points de dette supplémentaires par rapport à notre richesse nationale s'expliquent pour moitié par la dégradation de notre déficit, liée aux dépenses publiques que j'ai indiquées, mais pour moitié aussi, je tiens à le rappeler, par la diminution de notre richesse nationale, qui a baissé de 8,2 % en 2020. Cette hausse massive des dépenses publiques était le seul choix responsable pour faire face à la crise économique. Elle était nécessaire pour protéger nos salariés, éviter un chômage de masse et prévenir un tsunami de faillites d'entreprises. C'est le seul choix aussi qui permettra à l'économie française de rebondir vite et fort, dès cette année 2021, parce que nous aurons préservé nos entreprises, nos salariés, nos compétences, nos savoir-faire. Ma conviction est forte : en 2021, l'économie française repartira vite et fort. Les ressorts de l'économie française ne sont pas cassés. Nous avons subi une crise profonde, mais les fondamentaux de notre économie restent sains. Les entreprises restent prêtes à investir. Le plan de relance est bien calibré pour alimenter la croissance. Je le répète : en 2021, l'économie française repartira vite et fort. fort. Il nous appartient désormais, et c'est tout l'intérêt de ce débat, dont je remercie le Sénat, de faire en sorte que ce niveau d'endettement, qui sera l'héritage de la crise économique, ne devienne pas à long terme une vulnérabilité pour la France. C'est notre responsabilité à tous. La meilleure façon d'éviter que cette dette publique ne devienne une vulnérabilité pour la France, c'est de dire, de manière claire, sans aucune ambiguïté, que la France remboursera sa dette publique. Pour cela, il faut d'abord la stabiliser, puis engager sa réduction suivant une stratégie de remboursement sur laquelle je reviendrai. Je tiens à le préciser- ces propos rejoignent ce qu'a dit l'orateur précédent -, la France a en réalité deux dettes. La dette chronique est liée au niveau des dépenses publiques, qui est, je le rappelle, le plus élevé de tous les pays développés au monde.

près de 100 % du PIB à cause de cette dépense chronique qui caractérise l'économie française. Avec le Président de la République et l'ensemble de la majorité, nous avions réussi, pour la première fois depuis vingt ans, à réduire le déficit au-dessous de 3 % du PIB. Nous avions sorti la France de la procédure de déficit excessif. Nous avons tenu les comptes publics, diminué le taux de dépenses publiques

dans les technologies, les compétences, les savoir-faire, les chaînes de valeur qui permettront à la France demain de rester l'une des plus grandes puissances économiques de la planète. Cette dette choisie est une dette responsable et nécessaire quand les taux d'intérêt sont aussi bas et nous permettent

Je veux là aussi être très clair et profiter de ce débat pour rassurer nos compatriotes : la France n'a aucune difficulté à financer sa dette.

La dette a augmenté, mais tout le paradoxe est que, dans le même temps, la charge de la dette a nettement diminué parce que nous empruntons à des taux plus bas.

nous avons levé 290 milliards d'euros de dettes à moyen et long terme, soit près de 45 milliards d'euros de plus qu'en 2019. Pourtant, le taux moyen auquel nous avons emprunté ces 290 milliards d'euros est inférieur de 20 points de base au taux moyen de 2019. La récente émission d'une obligation à cinquante ans à un taux limité de 0,59 % atteste de la confiance des investisseurs dans la signature française,

Vous me direz que les taux d'intérêt- cela a été signalé par M. Bascher -, qui étaient de-0,30 % en début d'année, se sont rapprochés aujourd'hui de 0 %, avec un taux pour l'OAT à dix ans de-0,10 % hier soir. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude. Cette hausse est naturelle et maîtrisée. Elle est liée aux perspectives de reprise de l'activité économique, ... Il faut conclure, monsieur le ministre ! ... au nouveau plan de relance américain et au rebond de l'inflation qu'il peut susciter. Ce mouvement haussier est donc naturel et, je le redis, limité. La BCE a d'ailleurs assuré qu'elle maintiendrait des conditions de financement favorables.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Alors que notre taux d'endettement a bondi de 20 points en moins d'un an et qu'il dépasse désormais 120 % du PIB, une telle capacité à résorber la dette laisse rêveur. Mais comparaison n'est pas raison, et la situation en 2021 diffère largement de celle de l'après-1945, quand bien même nous déclarons la guerre au virus. L'économie doit repartir, et repartir vite, mais le pays n'est pas à reconstruire. La situation est aujourd'hui des plus singulières d'une part, la dette publique, en valeur absolue, n'a jamais été aussi élevée ; d'autre part, l'épargne privée, constituée pour une large part grâce aux mesures mises en place par le Gouvernement, n'a jamais été aussi On peut y voir un paradoxe historique. On peut aussi y voir une opportunité pour accélérer la relance sans dégrader davantage nos finances publiques. Si le Gouvernement ne dirige plus l'épargne des Français, et c'est heureux ainsi, il peut mettre en place des outils afin de l'orienter vers des investissements stratégiques.

Il y a la mauvaise manière, celle qui a été employée pendant des décennies : les impôts. Pour ma part, j'exclus toute augmentation d'impôts pour rembourser notre dette publique. Ce serait une erreur politique et une faute économique.

faut aussi, comme vous l'avez parfaitement indiqué, utiliser l'épargne des Français, qui auront constitué près de 200 milliards d'euros d'épargne d'ici à la fin de l'année. Nous voulons les inciter à transmettre plus facilement cette épargne à ceux qui pourraient la consommer. Je ferai des propositions au Premier ministre et au Président de la République en ce sens.

Enfin, la troisième manière de rembourser notre dette, c'est d'engager des réformes de structure. Nous avons commencé à le faire avec la réforme de l'assurance chômage. Vous connaissez également mes convictions concernant la réforme des retraites : j'ai toujours estimé qu'il fallait inciter les Français

je dirai qu'elle en a trois, même si je ne suis pas forcément d'accord avec votre caractérisation des deux premières. La troisième, c'est la dette écologique. Avec votre façon de compter,

Le « quoi qu'il en coûte » a permis à des millions d'entreprises et de Français de faire face à la crise sanitaire et économique. Rappelons-le, depuis le début de la crise, les mesures d'urgence ont représenté 106 milliards d'euros, soit 4,4 % du PIB. Au total, plus de 13 milliards d'euros ont été affectés aux mesures sanitaires, 62 milliards à la préservation de la main-d'oeuvre et au soutien aux revenus des ménages, 22 milliards d'euros à la liquidité des entreprises, et une enveloppe de 8 milliards d'euros a été spécifiquement fléchée vers les secteurs les plus touchés. Ce soutien indispensable a un coût. La dette française est ainsi passée de 98 % à près de 120 % du PIB. C'est un phénomène international, puisque le niveau de la dette publique et de développement économiques (OCDE). Face à une telle situation, les hypothèses et les débats autour de l'avenir de la dette se multiplient. Cependant, je crois que nous devons éviter de mettre tous les oeufs dans le même panier. Chacun doit pouvoir distinguer le cantonnement de l'annulation. L'annulation de la dette serait en effet une faute politique et un non-sens économique. Inutile, voire contreproductive, elle aurait conséquences sur la crédibilité financière de la France. L'hypothèse du cantonnement, quant à elle, demande sans doute une plus grande attention de notre part. D'ailleurs, avons-nous les moyens de cantonner la dette covid ? De la quantifier pour mieux l'isoler ? Et si cela est envisageable, qu'en est-il de son remboursement ? La France sait gérer sa dette sociale. Et elle savait le faire avant la crise de la covid. Avec la création de la Caisse en 1996, la dette sociale était passée de 260 milliards à 100 milliards d'euros en 2019, et il était prévu de l'apurer dès 2024. Entre-temps, la crise est passée par là. Elle a sans aucun doute modifié le calendrier.

sur le « quand », je redis que le rétablissement des finances publiques ne pourra être engagé que lorsque la crise sera derrière nous. Rien ne serait plus dommageable à la protection de notre économie que d'appuyer à la fois sur le frein et sur l'accélérateur.

Les conséquences de la crise de la covid-19 sur nos finances publiques sont inquiétantes : la dette publique pourrait atteindre plus de 120 % du PIB à la fin de l'année. La Commission européenne a réagi avec célérité au mois de mars 2020 en suspendant ce qui a longtemps été considéré comme une « sacro-sainte » règle le niveau maximal d'endettement à 60 % du PIB. Pourtant, ce seuil a été largement franchi sans que les marchés financiers s'affolent, grâce à l'action expansionniste de la Banque centrale européenne Les chiffres nous auraient horrifiés avant la crise. Mais, partout au sein de la zone euro, cette « ligne rouge » a été franchie, afin de profiter au maximum des marges de manoeuvre budgétaires et de relancer l'activité économique. telle dégradation de la situation de nos finances publiques doit être temporaire. Vous l'avez dit, le retour à la croissance devra nous permettre de rembourser la dette. J'entends de nombreuses propositions de modalités de remboursement dans le débat public qui méritent que le Parlement s'y attarde. Je pense en particulier au cantonnement de la dette covid, suggestion formulée par le Haut-Commissaire au plan. Mais ne devons-nous pas profiter de cette situation exceptionnelle pour réviser les règles européennes d'encadrement des finances publiques, qui ont révélé durant la crise leur obsolescence dans la mesure où elles empêchent d'investir pour notre avenir ?

sur la scène européenne, la priorité absolue est accordée à sa mise en oeuvre. Vous savez combien il a été difficile de convaincre l'ensemble des partenaires ; M. le ministre de l'économie pourrait en témoigner. Nous travaillons aujourd'hui avec la Commission. Nous échangeons sur les modalités de mise en oeuvre et de décaissement, pour évoquer les choses le plus clairement possible. Nous discutons de la préparation des différents plans de relance et du plan de résilience que chaque État doit présenter devant la Commission dans les prochaines semaines.

de ces mesures d'assistanat et de ces cadeaux fiscaux ou niches en tous genres, l'État n'est rien d'autre qu'une victime résignée des marchés financiers. Non seulement les ménages les plus aisés et les grandes entreprises bénéficient de politiques accommodantes, mais en plus, ils sont nos créanciers puisqu'ils détiennent des obligations d'État. Et vous le savez ! La parole est

quels que soient les gouvernements successifs, le message permanent envoyé aux Français était que nous devions contraindre nos dépenses publiques pour contenir notre dette sous peine de voir celle-ci devenir insoutenable. Aujourd'hui, alors que la dette vient d'augmenter de plus de 20 % en un an, comment s'étonner que nos concitoyens s'interrogent sur le remboursement à venir d'une dette née de la pandémie et, par ailleurs, parfaitement justifiée ? Comment s'étonner qu'ils ne comprennent pas qu'un taux d'endettement de 98 % du PIB ait pu être jugé inquiétant début 2020 et qu'un taux de 120 % soit parfaitement soutenable début 2021 ? Comment s'étonner qu'ils ne se préparent pas en payer le prix, thésaurisant quand ils le peuvent, d'autant plus quand le Gouvernement n'attend même pas la fin de la pandémie pour ressortir la réforme des retraites comme « la » solution au problème ? Nous le savons tous, le temps d'adaptation et de redécollage de notre économie est fixé par la politique monétaire de la BCE, et par rien d'autre. Sauf remontée brutale d'une inflation qui l'obligerait à modifier sa politique, la Banque centrale soulage l'État d'un éventuel risque de remontée des taux d'intérêt pour 25 % de sa dette, ce qui est un soutien considérable, sans doute pour de longues années. Cette fraction de dette ne coûte donc quasiment rien.

diminuer. Avant de se lancer dans une simple politique de rééquilibrage de nos comptes publics visant notamment à assurer dans le temps long la soutenabilité de la dette, ne faudrait-il pas poser

Comme vous l'avez indiqué, la politique budgétaire a pris depuis maintenant un peu plus d'un an le relais de la politique monétaire de la BCE. C'est ce qui nous

pour que des ingénieurs et des ouvriers qualifiés du secteur aéronautique, à Toulouse, en Occitanie et ailleurs, chez Airbus comme dans les PME sous-traitantes, puissent continuer à travailler, même s'il n'y a pas de commandes payées par de l'argent public. Ces compétences, ce sont des décennies d'investissement.

venu. Il viendra quand la croissance sera de retour et l'épidémie véritablement derrière nous. Si nous engageons trop rapidement le rétablissement des finances publiques, nous nous exposons à avoir une croissance plus faible et un chômage plus important. le pilotage du calendrier du rétablissement des finances publiques est un point-clé. Il est d'autant plus nécessaire d'avoir une stratégie claire ; nous venons de préciser la nôtre avec Olivier Dussopt.

Qui devra mettre la main à la poche ? Quand ? Comment ? Autant de questions qui les taraudent face à cette véritable bombe à retardement. À la délégation aux entreprises du Sénat, nous sommes tout particulièrement sollicités par les chefs d'entreprise : qu'ils soient dirigeants de grands groupes ou de PME, commerçants, artisans ou indépendants, tous sont inquiets pour l'avenir. Compte tenu de ce qu'ils disent, je pense que l'État n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir le tissu économique et social de notre pays. Ce Ce n'est que progressivement qu'il conviendra de diminuer les aides. Il faudra réduire graduellement l'importance de la perfusion, et non pas l'arracher brutalement. Malgré ce soutien, les défaillances d'entreprises sont encore devant nous. Monsieur le ministre, en avez-vous évalué l'effet économique et social, et le poids supplémentaire pour le budget de l'État ? Aujourd'hui, le Gouvernement donne le sentiment de naviguer à vue, sans un horizon clair. C'est un peu court, vous en conviendrez, pour donner aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin. Véritables semelles de plomb pour les entreprises, les impôts de production ont commencé à décroître. C'est heureux ! Leur niveau handicape gravement la compétitivité française. Mais l'État ne sera-t-il pas tenté de se rattraper, au risque de lever une tempête de ras-le-bol fiscal ? Les entreprises craignent la double peine : devoir rembourser à la fois leurs propres dettes, très alourdies par la crise, et celle de l'État les impôts

Monsieur le sénateur, je vous le redis avec beaucoup de clarté et de fermeté : j'exclus toute augmentation d'impôts,

partielle, seront maintenus tant que la crise touchera les secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture, du sport ou de l'événementiel. Je veux dire aux chefs d'entreprise concernés que nous ne retirerons pas brutalement ces dispositifs.

Et puis, il y a d'autres secteurs de l'économie qui ont déjà commencé à redémarrer fortement. Encore une fois, l'économie française va redémarrer vite et fort quand les contraintes sanitaires seront levées. Dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'agroalimentaire, dans beaucoup de secteurs de haute technologie, nous la confiance revenir et les investissements redémarrer. Nous voulons accompagner ces entreprises en mettant à leur disposition des prêts participatifs dont je préciserai les modalités jeudi matin. Ce sont de quasi-fonds propres. Ils permettront aux entreprises de se projeter dans l'avenir, d'investir et d'embaucher. Car j'ai une confiance totale dans la capacité de rebond de notre économie et de nos entrepreneurs.

La dette de notre pays est une préoccupation forte pour bon nombre de nos concitoyens. Au nom du groupe Union Centriste, je souhaite poser deux questions, qui sont aussi des propositions. Premièrement,

Le débat sur l'annulation de la dette nous conduit à rappeler aujourd'hui notre opposition au choix de l'exécutif d'imputer aux comptes sociaux le remboursement de cette dette covid. Le cantonnement de la dette, s'il a l'avantage de laisser penser que celle-ci est mise de côté, ne changera visiblement rien aux réformes que vous avez décidé de mettre en place. Il ne s'agira en fait que d'opérations de tuyauterie. Nous avons pourtant l'obligation d'augmenter dès maintenant les ressources de l'hôpital public, d'alimenter la cinquième branche que vous avez créée et d'améliorer le sort des salariés de tout le secteur sanitaire et social. Dans ce contexte, et avec comme objectif de protéger les comptes sociaux, envisagez-vous de dégager la sécurité sociale du remboursement de la dette covid ?

de la crise covid. Celle-ci nous paraît devoir être ainsi cantonnée pour permettre à l'Acoss de continuer à travailler de manière aussi autonome et sereine que possible. La dette sociale que nous voyons s'accumuler à l'occasion de la crise n'est pas liée à un désengagement de l'État.

du déficit pour l'année 2020, sachant que le maintien de l'activité à un niveau plus important que prévu nous a aussi permis de limiter la casse. Nous aurons certainement un déficit moins élevé que ce que nous craignions, même s'il restera particulièrement important.

largement et nettement votre affirmation sur la remise en cause du modèle social et des acquis sociaux. Enfin, la volonté de faire peur n'empêche pas la précision. Vous avez évoqué la réforme de l'assurance chômage : je suis désolé de vous dire que le déficit de l'Unédic n'a pas grand-chose à voir avec celui de la Cades ... La parole est à Mme Monique Lubin, pour la réplique.

Avant la crise, elle ne représentait que 11 % de la dette publique. Mécaniquement, elle a baissé et, aujourd'hui, elle doit se situer aux alentours de 8,5 %. On pourrait donc considérer que ce n'est pas vraiment un problème. Mais je me souviens qu'à l'automne 2017, au moment où l'État discutait des fameux contrats de Cahors, qui visaient à imposer aux plus grosses de nos collectivités locales- 327 de mémoire -une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement limitée à 1,2 % par an, le Gouvernement avait également eu l'idée de mettre en place une règle d'or renforcée qui aurait contraint ces mêmes collectivités locales en limitant leur capacité d'endettement.

Nous notons que la capacité de financement des sections d'investissement reste extrêmement importante, à plus de 31 milliards d'euros, tout comme le niveau global de trésorerie des collectivités, à plus de 48 milliards d'euros. Avec le maintien des dotations

la dette française s'élève à plus de 120 % du PIB, soit 2 700 milliards d'euros, dont on ne connaît pas exactement les détenteurs. En effet, les données ne permettent de dégager que des ordres de grandeur,

sur leur répartition catégorielle ou géographique. En avril 2019, selon les données du FMI, la part de la dette française des non-résidents serait détenue à 47 % par des investisseurs privés non bancaires, institutionnels ou non, et à 53 % par des institutions publiques et des banques étrangères. Les données issues de la même enquête de 2019 permettent d'identifier que les non-résidents non européens sont majoritaires, l'étude agrège dette publique et dette privée. La France est donc majoritairement endettée vis-à-vis de l'extérieur. Or un État souverain doit pouvoir disposer de photographies régulières de ses créanciers.

spéculatifs, mais aussi pour ajuster sa stratégie de financement et de remboursement. D'un point de vue juridique, aucun dispositif d'identification des porteurs de titres publics n'est prévu par la loi, à la différence

toutefois relativiser cette situation dans la mesure où la détention d'une part de la dette souveraine ne donne aucun droit à l'investisseur sur la conduite de la politique du Gouvernement ou la détermination des choix de la Nation.

Nous ferons tout ce qui pourra être fait dans les deux années restantes du quinquennat pour stabiliser et baisser la dette publique française. Croyez-moi, nous prendrons les décisions nécessaires

augmentation du nombre de chômeurs et d'entreprises en faillite, tout en sachant pertinemment que la crise est loin d'être terminée. Comment croire dès

Lavarde. En janvier 2020, la Commission européenne décidait de suspendre temporairement le pacte de stabilité et de croissance pour permettre aux États membres de lutter contre la pandémie de covid.

Les ministres des finances de l'Eurogroupe ont pour la plupart exprimé leur souhait de restaurer le pacte en 2021. Est-ce la position du gouvernement français ? En novembre 2019, le Président de la République, dans une interview accordée

Vous avez raison, madame la sénatrice, toutes les décisions que nous prenons s'inscrivent dans une perspective européenne. Avant même de parler d'indicateurs du pacte de stabilité et de croissance, je rappelle qu'il existe un plan de relance européen,

La parole est à M. Sébastien Meurant. Il n'y a pas d'argent magique, disait le Président de la République. Pourtant, la dette publique explose, conséquence de la lâcheté des gouvernements successifs qui ont délaissé depuis des décennies l'art difficile des choix politiques. Récemment, de beaux esprits se gargarisaient de vains espoirs. « Il ne sera pas nécessaire de rembourser la dette », nous disaient-ils, « ou, même s'il faut la rembourser, les taux négatifs ou faibles rendront l'opération indolore

Là encore, revenons aux fondamentaux. Un revenu est toujours lié à un travail, soit un travail actuel rémunéré, soit un travail ancien qui a permis d'accumuler un capital. Nous vivons dans un monde qui semble totalement virtuel, où l'investissement privé est déconnecté de l'épargne, l'investissement public déconnecté de l'effort fiscal, le revenu déconnecté du travail ! À l'heure où les mots « développement durable » sont sur toutes les lèvres, nous pouvons dire, sans risque d'être contredit, que ce modèle de développement ne l'est pas. Il est temps, mes chers collègues, de revenir à la raison et de réapprendre à gérer, comme l'on disait naguère, « en bon père de famille ». Le monde réel est brutal. Si nous ne revenons pas au bon sens, d'autres nous y contraindront. Cessons de croire qu'une chose ne coûte rien sous prétexte que « c'est l'État qui paye », comme disait M. Hollande, ou que l'on peut mener des politiques « quoi qu'il en coûte », comme le prétend aujourd'hui son brillant disciple. Monsieur le ministre, vous n'avez pas la maîtrise de la politique monétaire. Que ferez-vous si les taux repartent à la hausse ?

-et débrancher progressivement les dispositifs d'aide d'urgence pour revenir à un niveau plus soutenable de dépenses publiques. Une fois que nous aurons fait cela et que nous serons sortis de cet épisode de crise

et de gestion du stock de dette nous étions relativement confiants, parce que notre signature est garantie et reconnue et parce que la politique monétaire est bien orientée.

nous n'avons jamais réduit le poids de la dette, même quand nous avions 1,5 % de croissance, parce que nous sommes incapables de diminuer les dépenses de l'État qui vous sont chères,

mais nous avons maintenu cette politique avec beaucoup de constance et de lisibilité. Nous nous étions engagés à baisser le taux de l'impôt sur les sociétés à 25 % en 2022 pour revenir dans la moyenne européenne ; il sera ramené à 25 % en 2022. Nous nous étions engagés à supprimer la taxe d'habitation ; elle sera supprimée.

c'est l'émission de dette commune voulue par la Chancelière allemande, Angela Merkel, et le Président de la République française, Emmanuel Macron. Je vous en supplie : pour l'intérêt du débat, revenons aux réalités et écartons les affabulations Monsieur le ministre, vous n'avez pas bien compris mes propos. Je vous ai dit que vous aviez baissé les impôts en ayant recours à de la dette supplémentaire. Ce recours systématique

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, il me revient de conclure, pour aujourd'hui, ce débat sur la dette publique demandé par le groupe Les Républicains. Beaucoup a été dit et je souhaiterais profiter du temps qui m'est imparti pour proposer quelques grands principes qui pourraient guider notre stratégie budgétaire à venir. Au terme de ce débat, il me semble que l'on peut s'accorder sur le fait qu'il existe deux motifs légitimes d'endettement. Le premier, de s'endetter pour investir dans l'avenir. Lorsque l'État finance à crédit un projet d'investissement, dont le rendement est supérieur à son coût de financement, il fait une bonne opération. Le second motif légitime d'endettement, c'est de soutenir le tissu productif en cas de choc économique. La politique budgétaire doit alors être mobilisée pour atténuer ce choc et éviter que la croissance ne soit trop durablement pénalisée. Quel regard porter sur la dette française au regard de cette grille de lecture ? Pour reprendre la distinction de Mario Draghi entre la « bonne » et la « mauvaise » dette, il me semble qu'un large consensus existe pour considérer que la dette d'avant-crise était en grande partie de la « mauvaise » dette. Si les pouvoirs publics ont toujours soutenu l'économie en phase de ralentissement, une réelle volonté de retrouver des marges de manoeuvre budgétaires en sortie de crise a manqué. Ainsi, l'actuelle majorité n'a pas profité de l'embellie conjoncturelle du début de quinquennat pour réduire notre déficit structurel. Je vous épargnerai la comparaison, cruelle, avec l'Allemagne ... En outre, la hausse continue de l'endettement depuis les années 1980 ne s'est pas accompagnée d'un effort particulier de dépenses utiles à la croissance. En réalité, l'endettement a simplement financé des dépenses courantes. Si la dette pré-covid était donc de la « mauvaise » dette, la dette covid me paraît constituer, à l'inverse, de la « bonne » dette. En effet, si l'État n'avait pas soutenu les entreprises et les ménages, les faillites auraient atteint des niveaux jamais observés, ce qui aurait grevé les recettes publiques en sortie de crise au risque de compromettre notre capacité de remboursement. Ce soutien massif a été d'autant plus opportun que la dette covid a été contractée, vous le savez, à taux négatif : elle ne commencera donc à nous coûter que lorsqu'elle sera refinancée sur les marchés, soit dans un peu moins de dix ans en moyenne. Dès lors, gardons-nous de débats inutiles sur la nécessité de cantonner ou d'annuler cette dette qui demeurera encore longtemps « gratuite » pour la France. Si ce diagnostic est largement partagé, les avis sont plus divergents concernant l'avenir de notre stratégie budgétaire. Il faut à mon avis distinguer deux temps. Le premier temps est celui de la crise qui, malheureusement, n'est toujours pas terminée. Soutenir temporairement le tissu productif et les ménages à court terme reste la bonne stratégie sur le plan économique et budgétaire. Il ne faut pas chercher à redresser les comptes publics avant que l'économie retrouve ses capacités de production au risque, sinon, de casser l'appareil productif, puis la reprise, ce qui nous amène en fait à 2023. En cas d'aggravation de la crise, il ne faudrait pas hésiter à réviser encore à la hausse les mesures de soutien et de relance. Une fois la crise surmontée viendra le second temps, celui du redressement des comptes publics. Sur ce plan, l'objectif du prochain quinquennat devrait être de stabiliser l'endettement pour rassurer les marchés. Avec une croissance nominale de 2,5 % et un endettement de 120 % du PIB, suppose de ramener le déficit autour de 3 % du PIB, alors que le déficit structurel devrait être de l'ordre de 5 % à 5,5 % en sortie de crise. Cela représentera un effort d'économies significatif de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros.

Ensuite, il faut dès maintenant réfléchir aux réformes structurelles susceptibles d'entraîner des économies, car elles mettent toujours du temps pour produire leurs effets budgétaires.

Tirons les enseignements du passé ! S'il faut réaliser des économies, en traquant les dépenses courantes inefficaces, il ne faut pas pour autant sabrer dans les investissements publics. Permettez-moi enfin d'insister sur la nécessité d'investir pour la transition écologique.

conclure. Ainsi, les services de l'Insee ont récemment évalué notre dette climatique à 150 % du PIB. Cela donne la mesure des efforts qui seront à entreprendre en la matière

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Républicains a décidé d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat « Comment construire plus et mieux en France ? » après celui qui avait été organisé sur le logement en juin dernier, car les craintes que nous exprimions au sortir du premier confinement sont devenues réalité. La crise sanitaire a entraîné un approfondissement de la crise du logement et de la construction. Les chiffres de 2020 sont alarmants. Environ 90 000 logements sociaux ont été agréés ; il y en avait plus de 120 000 en 2016. Tous logements confondus, on compte 73 500 permis de construire de moins en

Je vous propose d'en analyser les causes avant d'esquisser des pistes de solutions qui seront approfondies au cours du débat. Tout d'abord, quelles sont les causes de cette dramatique chute de la construction ? À écouter le Gouvernement, il y aurait deux coupables : les maires, frileux pour construire en raison des élections municipales, et le virus.

ne sont donc pas si coupables ... Que dire du virus ? Il est bien évident qu'il a grippé la machine, mais à y regarder de plus près, si les courbes ont piqué du nez en 2020, elles fléchissent depuis 2017. Ainsi, derrière la conjoncture très difficile de l'année 2020, il y a des causes structurelles qui sont liées à la politique du Gouvernement. Tous les acteurs du logement social le disent : ce sont bien les ponctions faites sur les bailleurs sociaux et sur Action Logement qui sont la cause profonde de la chute très inquiétante du nombre de logements sociaux

En réalité, le Gouvernement a mené jusqu'à présent une politique malthusienne de décroissance et d'économie budgétaire : « la politique du logement coûterait trop cher en France et serait inefficace, puisqu'il n'y aurait d'ailleurs pas de crise du logement mieux vaudrait rénover que construire » ; « il n'y aurait plus besoin de financements publics, car les taux sont bas et les institutionnels prêts à investir ». Voilà, au fil des rapports ou des notes administratives, la petite musique que l'on entend depuis quatre ans et qui sape peu à peu la dynamique de la construction et du logement social. C'est un fait ! Selon le rapport annuel du compte du logement publié fin 2020 par votre ministère, les aides au logement ont reculé : elles représentaient

Parallèlement, le mal-logement n'a jamais été aussi important dans notre pays. Selon la Fondation Abbé Pierre, il frapperait plus de 14 millions d'habitants, ainsi privés de logement personnel ou vivant dans des conditions difficiles. On sait par ailleurs qu'il y a plus de 2 millions de demandes de logements sociaux pour 450 000 attributions annuelles. Enfin, la population française croît et les évolutions sociales favorisent la décohabitation. La demande de logements est donc soutenue. La crise du logement est réelle dans de nombreux territoires, elle n'est pas une lubie. Construire plus et mieux n'est pas une option, c'est une absolue nécessité Mais comment y parvenir ? Je voudrais proposer trois pistes : aider, libérer, densifier. Aider tout d'abord. Je l'ai dit, la réduction des capacités d'investissement des bailleurs est l'une des causes structurelles

viennent confirmer ce besoin. Aider les bailleurs et les promoteurs est certes important, mais aider les maires est tout aussi nécessaire. Les exonérations de taxes locales non compensées par l'État sont devenues un obstacle majeur au développement du logement social. Pour un maire, il peut être plus raisonnable de payer des pénalités que de construire. Sur 500 millions d'euros de dégrèvements, seuls 16 millions sont compensés ! Comment financer la viabilisation des terrains, les écoles, les équipements et les transports dans ces conditions ? Deuxième axe : libérer. Les maires, comme les promoteurs et les bailleurs privés, se plaignent des contraintes qui pèsent sur eux. Au sortir de la crise, après avoir écouté promoteurs, architectes, aménageurs et élus, j'avais proposé un Ségur de la simplification de l'urbanisme, non pas comme une grand-messe, mais comme un exercice concret réunissant praticiens et juristes pour simplifier l'acte de construire et réduire enfin les délais et les coûts.

pourtant moins cher, et de créer un statut du bailleur privé vu non pas comme un rentier, mais comme un entrepreneur en logement. Troisième axe : densifier. Nous le savons, c'est la clé pour construire plus et mieux et pour limiter les conséquences néfastes de l'étalement urbain, mais, nous le savons tout autant, la densité fait peur et rencontre l'opposition de nombreux citoyens. Il faut la faire accepter. Je suis convaincue que c'est possible si l'on aide les maires bâtisseurs et si l'on propose de beaux projets qualitatifs correspondant aux demandes sociales et de véritables projets urbains, où densité rime avec solidarité et proximité des services. Le concept de « ville du quart d'heure de l'urbaniste Carlos Moreno a rencontré le succès médiatique. Peu importe le terme, relevons le défi de concevoir des villes pour le XXI siècle ! Construire plus et mieux est vital pour loger tous les Français. C'est également vital pour notre économie. Mais plus largement, dans cette période de crise et de doute, nous avons besoin d'imaginer un futur meilleur. Construire est un acte d'espérance et de foi dans l'avenir. C'est un bien essentiel.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, en engageant ce débat sur le thème « Comment construire plus et mieux en France ? », je voudrais tout d'abord saluer l'engagement et le travail du Sénat sur les questions liées aux politiques du logement.

Cette question est bien au coeur de l'action du Gouvernement, qui n'oppose pas rénovation et construction, et des mesures importantes ont été prises pour répondre à la crise exceptionnelle que nous traversons.

En prenant uniquement les années 2018 et 2019, les chiffres de mises en chantier, comme ceux des permis de construire, sont supérieurs à ceux de la décennie précédente. Nous étions donc sur une tendance positive, mais cette dynamique a effectivement été freinée en 2020,

Donc non, la construction n'a été oubliée ni par la relance ni par l'État ! Tout d'abord, un effort particulier est déployé pour le logement social. Deux millions de Français sont actuellement en attente d'accéder à un logement social. La crise que nous traversons accentue cette demande de la part de nos concitoyens. J'ai donc décidé de proposer à tous les acteurs du secteur de faire de 2021 et 2022 des années de mobilisation générale pour la relance de la construction de logements sociaux, en allant nettement au-delà de l'objectif annuel de 110 000 logements sociaux qui était atteint avant 2020.

Concrètement, en 2021, la Caisse des dépôts va mobiliser 300 millions d'euros supplémentaires pour souscrire des titres participatifs auprès des bailleurs sociaux. Sur la période 2021-2022, CDC Habitat s'engage à produire 42 000 logements sociaux nouveaux, soit une augmentation de 50 % de sa production annuelle par rapport à 2020. Action Logement mobilisera pour sa part, dans le cadre de la convention que nous venons de signer, 500 millions d'euros de subventions exceptionnelles pour le logement social et Action Logement Immobilier a prévu de développer plus de 70 000 logements sociaux nouveaux sur deux ans.

C'est la raison pour laquelle, dans le plan de relance, le Gouvernement mobilise 650 millions d'euros pour la viabilisation des friches et la densification urbaine. Dans ce cadre,

Construire plus et mieux nécessite de simplifier les procédures. Plusieurs actions ont été entreprises en ce sens, notamment la mise en oeuvre de la dématérialisation des documents d'urbanisme, ainsi que la suppression de l'agrément pour le logement locatif intermédiaire.

Nous avons par ailleurs supprimé l'agrément préalable des opérations de logements intermédiaires- cette mesure a été votée par le Sénat -et j'ai pris un arrêté, à l'automne, pour simplifier drastiquement le dossier d'agrément des logements sociaux. L'État a donc mis en place les moyens et les dispositifs nécessaires au rebond en 2021 et 2022, mais il est vrai qu'en matière de construction, comme pour de nombreuses politiques, l'État ne peut pas faire seul et les élus locaux jouent un rôle important. Nous le savons tous ici, ce sont les maires et les élus intercommunaux qui déterminent les règles d'urbanisme et délivrent les permis de construire. Les professionnels nous alertent aujourd'hui sur la multiplication des cas de blocage de permis de construire, pourtant conformes aux règles d'urbanisme et au plan local d'urbanisme (PLU), et sur la remise en cause de projets de logements déjà lancés. Le véritable danger, c'est de refuser d'accueillir des populations nouvelles, de ne répondre qu'aux besoins des habitants en place et, ce faisant, de refuser de répondre aux besoins des jeunes qui décohabitent, des familles qui déménagent ou des personnes qui connaissent une mobilité professionnelle et ont besoin d'un nouveau logement.

C'est pourquoi la mobilisation collective est importante et revêt une dimension politique. J'ai ainsi signé en novembre dernier, avec toutes les associations de collectivités territoriales, un pacte pour la relance de la construction durable, et je salue l'engagement de certaines villes, comme Dijon, ... Au hasard ! ... Les préfets, avec lesquels j'étais encore ce matin en réunion, les sous-préfets à la relance et l'ensemble des services de l'État sont aux côtés des territoires et missionnés pour soutenir cette mobilisation collective, mettre du liant avec les acteurs locaux et favoriser, chaque fois que c'est possible, la mise en oeuvre des projets. Enfin, il faut projeter vers l'avenir une vision de la construction et du logement dans une logique d'aménagement du territoire. Concernant le volet social tout d'abord, il faut continuer à travailler sur la loi relative à la solidarité et au renouvellement qui permettra de porter cet objectif ambitieux tout en trouvant les souplesses nécessaires, est inscrite dans le projet de loi dit « 4D » qui vient d'être soumis au Conseil d'État. Nous souhaitons maintenir l'exigence mais tenir compte des situations locales, en nous appuyant sur les propositions faites par la commission SRU présidée par Thierry Repentin ont recueilli l'avis favorable de l'ensemble des parties prenantes et feront l'objet d'une transcription législative. Mais construire mieux, c'est aussi construire, dans une vision d'aménagement du territoire, des logements confortables et performants sur le plan environnemental. Pour favoriser l'aménagement du territoire, il faut trouver la manière de proposer des projets de densité suffisante qui permettent de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols et d'inclure des services, tout en restant désirables. C'est pourquoi, dans une démarche que j'appelle « Habiter la France de demain

puisqu'il est responsable de 19 % des émissions nationales de dioxyde de carbone et de 60 % des tonnes de déchets produits en France. Des mesures fortes et ambitieuses sont aujourd'hui indispensables pour atteindre l'objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Bien sûr, nous devons continuer à construire plus. Je souhaite concentrer mon propos sur l'écoconstruction, encore bien trop marginale alors que ses bénéfices sont multiples- écologiques, locaux ... -et qu'elle présente une utilité sociale forte, car elle permet de lutter efficacement contre la précarité énergétique.

Un mur porteur en briques de terre cuite consomme quatre fois moins d'énergie grise qu'un mur en béton armé. Certains de ces biomatériaux permettent de stocker des quantités de carbone très importantes : un mètre cube de bois massif mis en oeuvre sur chantier stocke 460 kilogrammes de CO2, alors qu'un mètre cube de béton en émet l'équivalent le gain carbone est donc de quasiment une tonne de CO2 par mètre cube. Ces logements passifs procurent un confort thermique inégalable. Leur degré d'hygrométrie et leur inertie permettent de rafraîchir l'air ambiant, et donc de se passer de climatisation. lorsque ces habitations doivent être déconstruites, elles retournent à la terre, d'où elles viennent, en produisant peu de déchets puisque la majeure partie de ces matériaux est biodégradable. Il s'agit donc d'un cercle vertueux. Madame la ministre, allez-vous lever les obstacles pour créer de véritables filières locales de l'écoconstruction,

Cette nouvelle réglementation, dont les derniers ajustements ont été présentés il y a une petite dizaine de jours, porte une ambition extrêmement forte qui soutiendra le développement des matériaux biosourcés dans la construction. a trois objectifs principaux : la sobriété énergétique, la diminution de l'impact carbone dans la construction des bâtiments, et enfin la fraîcheur en cas de fortes chaleurs l'été.

au cycle de la construction lui-même. L'obligation de réduire progressivement jusqu'à 30 % les émissions de gaz à effet de serre lors du process de construction, tout en garantissant la possibilité de mixité des matériaux, favorisera le recours à des matériaux biosourcés tels que le bois

climatique. Cette réglementation entrera en vigueur progressivement, dès le 1 janvier 2022 pour la baisse de la consommation,

Ainsi, avec le soutien financier de l'État à hauteur de 1,5 milliard d'euros, 250 000 logements sociaux pourraient être construits dans les deux ans à venir. Si nous pouvons nous satisfaire de cet objectif ambitieux, mon interrogation porte sur la part de logements sociaux prévus en outre-mer. Comme vous le savez, ces territoires font face à des besoins grandissants liés aux flux migratoires, aux mutations culturelles telles que la préférence pour l'habitat individuel, au phénomène de la décohabitation, à la prégnance de la précarité et surtout

ouvrant droit à des logements très sociaux, contre 29 % en métropole. Madame la ministre, sur les 250 000 logements sociaux que vous prévoyez de construire, quelle sera la part accordée aux territoires ultramarins, qui font également face à une pénurie de logements sociaux ? La parole

L'État s'engage et accompagne particulièrement les territoires d'outre-mer sur ces questions de logement et d'aménagement. Je souhaite souligner la création récente des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, qui ont pour priorité de produire des terrains aménagés nécessaires au développement de l'offre de logements et d'équipements dont ces territoires ont besoin de façon urgente. La production et la réhabilitation de logements sociaux sont financées par la ligne budgétaire unique sur le programme 123 du ministère des outre-mer à hauteur d'environ 10 000 logements par an- des logements sociaux, mais aussi des logements neufs relevant de l'accession sociale. Malgré la crise, la consommation de cette ligne, qui a atteint 218 millions d'euros en 2020, est en augmentation de 30 millions d'euros par rapport à 2019, et pour 2021, les crédits, de nouveau en nette hausse, s'élèvent à plus de 240 millions Une dynamique importante a donc pu être maintenue en 2020, alors même que le niveau d'agrément connaissait une chute en métropole. Il faut bien sûr veiller à maintenir cette dynamique en 2021

Comme vous le savez, ces objectifs quantitatifs précis sont donnés territoire par territoire dans le cadre des plans de logement outre-mer. Le plan d'investissement volontaire d'Action Logement, qui prévoit 1,5 milliard d'euros consacrés au logement en outre-mer, s'inscrit également dans cette territorialisation.

Alors que la crise du covid pèse toujours sur notre quotidien, il semble intéressant d'évoquer la construction de logements à la lumière des effets de la crise sanitaire sur ce secteur. Cette crise et le confinement qui l'a accompagnée, qu'il soit total ou partiel, ont d'autant plus révélé les défauts des logements que ceux-ci ont dû accueillir des fonctions inhabituelles. Il nous a fallu travailler à la maison, y faire l'école ou encore y pratiquer une activité sportive. La période actuelle a ainsi révélé la nécessité d'habiter des logements susceptibles de répondre à différents usages selon l'évolution des mesures adoptées pour limiter la propagation du virus. Le logement est devenu plus que le logement. De ce fait, des questions se posent. Si cette tendance devait durer et se confirmer dans le temps, l'habitat devrait être réinventé

En ces temps où nos mobilités sont limitées à l'extrême et nombre de nos activités empêchées, l'espace privé a en effet pris une importance inédite. C'est potentiellement tout notre rapport au logement et à son environnement immédiat qui aura été modifié par cette crise. La société dans son ensemble va devoir penser à l'après-crise pour répondre à ces attentes légitimes. du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, « nous ne pouvons plus imaginer des logements obsolètes avant d'être construits ». Comment allons-nous construire après ? Aux impératifs écologiques s'ajoute aujourd'hui une évolution des modes de vie et des besoins de la population qui est susceptible de perdurer, mais cette évolution des logements aura un coût comment créer des logements plus grands, plus confortables, dotés d'espaces extérieurs plus verts, tout cela à un coût supportable par les ménages et sans aggraver l'étalement urbain ? Madame la ministre, pouvez-vous préciser les attentes du Gouvernement quant au référentiel sur la qualité du logement en cours d'étude ?

ont été complètement oubliées. Face à cette situation, j'ai choisi de mandater de façon précise un architecte, François Leclercq, et un aménageur, Laurent Girometti,

L'objectif est de produire un référentiel simple qui permettra aux professionnels de se mettre d'accord sur le niveau de qualité du logement et sur la manière d'y parvenir. Ce référentiel n'a pas vocation à être une nouvelle norme, mais plutôt un point de repère commun

loi ALUR, visait à juste titre à réglementer l'urbanisme périurbain galopant qui détruisait les territoires ruraux de proximité. Mais elle a, en même temps, totalement bloqué l'urbanisation des territoires ruraux.

En outre, l'implantation très disparate des bailleurs sociaux, qui interviennent encore trop souvent en ordre dispersé, ne permet pas d'établir une stratégie coordonnée. Ce point a été souligné par la Cour des comptes, qui a suggéré une restructuration. Ces défis complexes doivent nous conduire à repenser l'intervention de la puissance publique en la matière sur ces territoires. Ainsi, compte tenu des spécificités des outre-mer, il faut territorialiser davantage la politique du logement, qui a besoin d'un pilotage clair, efficace et inscrit dans la durée. L'intervention de tous les acteurs du logement doit être coordonnée, en y associant davantage les collectivités locales. d'une meilleure lisibilité des critères de répartition et des réaffectations des crédits de la ligne budgétaire unique (LBU), la généralisation des plateformes d'ingénierie publique au niveau local doit être poursuivie et amplifiée. Étant donné le faible niveau de revenus des ménages ultramarins, le logement locatif très social doit être davantage priorisé. Face à ces constats, madame la ministre, et compte tenu du fait que le plan logement outre-mer 2015-2019 a été un semi-échec,

Le plan logement outre-mer 2019-2022, signé le 2 décembre 2019, constitue la base de notre action. Ce plan est très opérationnel et comporte de nombreuses mesures- 177 précisément -organisées selon quatre axes : la connaissance des besoins l'adaptation de l'offre aux territoires ; la maîtrise des coûts de construction et de réhabilitation ; la mobilisation du foncier et l'aménagement. Pour ce qui concerne la construction, les objectifs quantitatifs sont donnés territoire par territoire dans le cadre de plans territoriaux, donc au plus près des acteurs locaux.

prévoit notamment l'adaptation locale des documents techniques, le développement de filières de produits de construction locaux, l'installation d'organismes certificateurs outre-mer

2021 et 2022. Or, en l'état actuel des choses, vous n'avez strictement aucune chance d'y parvenir ! La première raison, rappelée par Marie-Noëlle Lienemann, est que ce sont les maires qui délivrent les permis de construire.

je tiens à saluer. Si nous n'avions pas trouvé ces moyens d'investissement, vous nous auriez dit : « Vous avez un objectif, mais pas de crédit pour investir dans le logement social : comment voulez-vous y arriver ? Il n'y aura pas d'investissement possible !

vous aurez perdu une année parce que tant que les maires n'auront pas la certitude d'une corrélation entre l'augmentation « tendancielle » de leurs ressources pour financer les équipements publics et le nombre de logements construits, les projets

tant quantitatif que qualitatif. D'une part, il faut construire plus pour répondre à la demande croissante de logements ; d'autre part, il faut construire mieux pour composer avec les nécessaires exigences environnementales. La loi ÉLAN a été porteuse- pour ne pas dire prometteuse -de simplifications

Il s'agit, au contraire, de simplifier celles qui existent et de les rendre compatibles entre elles pour construire davantage et plus vite, tout en répondant mieux aux enjeux climatiques. Par exemple, la RE2020, dont les arbitrages viennent tout juste d'être rendus publics, constitue un pari sur l'avenir. En effet, certaines exigences fixées essentiellement à l'horizon de 2028 à 2031 ne sont pas atteignables avec les technologies actuelles. Non seulement elles nécessitent de nouveaux process, de nouveaux matériaux et de nouvelles façons de faire, mais elles demandent également des adaptations très fortes de tous les métiers du bâtiment qu'il faut accompagner. Madame la ministre, que compte faire le Gouvernement pour simplifier les normes de la construction et pour accélérer les procédures d'urbanisme ?

Je citais précédemment la dématérialisation des autorisations d'urbanisme qui représente un progrès considérable, à la fois, pour les porteurs de projets, pour tous les services instructeurs et pour la liaison entre les services instructeurs des collectivités et les services de l'État qui sont saisis. Cette dématérialisation sera opérationnelle au 1 janvier prochain. Elle nécessite que l'État conduise un chantier d'envergure pour que les outils soient disponibles et puissent être choisis sous différents modèles par les collectivités. Je crois que ce sera un progrès.

Les différents jalons ont été placés en 2022, 2025, 2028 et 2031. L'ambition sur la construction elle-même est très progressive. Les filières industrielles sont respectées puisque nous avons veillé à préserver

Cette méthode est un levier déterminant pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone et pour lutter efficacement contre les changements climatiques. La transition vers une construction plus sobre bouleverse toutefois les méthodes des entreprises de la filière du bâtiment et de la construction,

pour tenir ces engagements, il faut un saut technologique et il est urgent d'investir dans l'outil de transformation industrielle, notamment du secteur bois qui ne bénéficie à ce jour ni du plan de relance ni du plan décarbonation.

la construction bois offre effectivement une formidable transformation en perspective pour le secteur. Elle représente une opportunité nationale, à la fois forestière, industrielle et territoriale. Elle constitue aussi un des leviers importants pour atteindre notre trajectoire climatique.

de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % donne toute sa place à la construction bois et aux matériaux biosourcés. Je vous rejoins sur le fait qu'il faut maintenant accompagner nos filières industrielles ; c'est une préoccupation que nous partageons avec Julien Denormandie et Agnès Pannier-Runacher. Nous sommes pour l'instant en retard, non seulement dans le segment du CLT (), matériau principal qui permet de construire des structures, mais aussi plus globalement en matière d'innovation sur les différents matériaux.

doté de 20 millions d'euros, pour soutenir des projets innovants favorisant la mixité des matériaux, dans le cadre du PIA4. Nous ouvrirons prochainement, avec Julien Denormandie et Agnès Pannier-Runacher, un deuxième appel à manifestation d'intérêt centré sur la filière bois, pour faciliter son industrialisation et un développement

je le dis souvent, l'idée du logement social c'est le logement pour tous ! Aussi, madame la ministre, je vous remercie d'avoir récemment rappelé que 70 % des Français sont éligibles à un logement social. Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans les défis qui attendent la société, y compris dans la relance économique à venir et pour permettre à la France de respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Prenons l'exemple, madame la ministre, d'un office HLM gardois que je connais bien pour l'avoir présidé pendant dix-sept ans. Alors que ses recettes locatives s'élèvent à 60 millions d'euros par an, l'impact de la RLS est de 6 millions d'euros. Malgré les efforts de gestion qui ont été accomplis et qui se poursuivent, cette perte de ressources financières entraîne une baisse des investissements de plus de 20 % au niveau des constructions neuves.

le rôle des commissions intercommunales d'attribution dans le projet de loi 4D qui sera prochainement présenté en conseil des ministres, puis examiné par votre assemblée. Pour répondre précisément à votre question sur la RLS,

que les bailleurs ont de nouveau les capacités financières pour atteindre des objectifs de production et de rénovation. Comme je vous le disais, nous avons pris de nouvelles mesures de soutien, en consacrant 500 millions d'euros de crédits du plan de relance à la rénovation des logements sociaux et 1,1 milliard d'euros au FNAP pour 2021 et 2022.

Les maires ont bon dos ! S'ils sont de plus en plus prudents sur l'octroi des permis de construire, c'est que depuis 2017, en particulier du fait de la loi ÉLAN, l'acte de construire est devenu un véritable parcours du combattant.

Ces maires que vous incriminez, il faut créer pour eux des incitations financières et réduire leurs contraintes administratives afin qu'ils octroient de nouveaux permis de construire. Bien évidemment, si l'on veut développer le logement social, il faut compenser largement l'exonération de TFPB, comme l'a dit très justement Marie-Noëlle Lienemann.

L'État fixe le cadre réglementaire, les normes d'urbanisme et les incitations fiscales. Les collectivités locales définissent ensuite les ambitions, les zones d'aménagement, les projets urbains, la construction et la capacité à façonner la ville. De nombreux maires l'ont fait au fil des années.

On constate pourtant à cet égard une différence de traitement entre les métropoles et les communes rurales, ces dernières connaissant de plus grandes difficultés à construire en raison de plans d'urbanisme restrictifs.

Il me semble donc indispensable d'apporter une réponse différenciée aux communes, notamment pour favoriser davantage celles qui n'ont pas connu de consommation de foncier excessive au cours des dernières années, et d'assouplir en conséquence les règles d'urbanisme qui les contraignent.

Il est en effet possible de bien construire, donc de construire mieux, dans les communes rurales. Les exemples de bâti peu consommateur de foncier, où la biodiversité est préservée, sont multiples : j'en connais dans mon département de la Haute-Vienne,

Construire plus, mais surtout mieux, et donner pour ce faire davantage de souplesse aux communes, telle est la stratégie essentielle à mettre en place si nous voulons pouvoir accueillir les populations urbaines qui envisagent, de plus en plus, de s'installer en zone rurale. C'est l'un des rares phénomènes positifs causés par la pandémie. Ne manquons pas cette occasion unique pour nos territoires, faute d'une meilleure politique de l'urbanisme ! Nous pourrons accélérer l'aménagement du territoire, développer des infrastructures de mobilité

La crise de la covid incite un certain nombre de nos concitoyens à s'interroger sur leur lieu de vie et, potentiellement, à sortir des grandes villes et des métropoles pour aller s'installer dans des territoires plus ruraux. C'est évidemment une chance pour ces territoires, qui doivent être en capacité d'accueillir ces populations. d'accueillir ces populations. Pour cela, il faut continuer à intensifier les politiques de rénovation et de réhabilitation des bâtiments déjà construits. C'est l'objectif des opérations de revitalisation des territoires (ORT) et des partenariats d'aménagement. Les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement sont à la manoeuvre, en première ligne, pour accompagner

qu'avec les collectivités territoriales. Dans la loi Climat et Résilience, nous fixons un objectif relativement modéré d'une réduction de l'artificialisation nette de 50 % dans les dix prochaines années.

Systématiquement, la responsabilité des élus locaux est remise en cause, alors que leur sensibilité aux questions de l'urbanisme intégré, de la consommation frugale des terrains, et de la qualité durable et économe du bâti est avérée.

Madame la ministre, seriez-vous prête à mettre en place, comme en Angleterre, un permis déclaratif sous la responsabilité du maire et d'un architecte DPLG, partout où des permis similaires ont déjà été autorisés, ou bien là où aucune difficulté particulière n'est patente ?

à l'échelon pertinent, qui est celui de l'agglomération ou de l'EPCI. Pour accompagner les EPCI dans le déploiement de ces nouveaux outils, les services de mon ministère ont mené un tour de France des PLUi Ils poursuivent ce travail pour recenser les SCoT et les PLUi exemplaires et partager ces bonnes pratiques. Fin 2020, on comptait 476 PLUi couvrant la totalité du territoire d'un EPCI déjà approuvés ou en cours ; 235 PLUi dits « sectoriels » sont également approuvés ou en cours d'approbation, soit environ 700 PLUi au total. Ce mouvement de planification a vocation à s'accélérer. En ce qui concerne les simplifications,

les permis de construire, lorsque ceux-ci sont conformes au PLU ou au PLUi. On sait en effet que, aujourd'hui, la majeure partie des permis déposés, qui sont conformes au PLU ou au PLUi, notamment en hauteur, sont systématiquement renégociés à la baisse par les élus, qui demandent que l'on remplace des constructions de

Nous le faisons non seulement des aides, là encore en partenariat avec Action Logement, pour l'adaptation des logements au vieillissement- ce sont des actions très concrètes comme le changement de baignoires en douches, par exemple -, mais aussi dans le cadre du développement de l'habitat inclusif.

Je vais prendre l'exemple d'une commune du Gard, Milhaud. La justice administrative a annulé une décision du maire de cette ville, qui refusait un raccordement au réseau électrique. Ce refus était pourtant motivé par le fait que les élus ne souhaitaient pas laisser s'installer des logements précaires

depuis, le propriétaire s'est fait livrer plusieurs Algeco. Cerise sur le gâteau, la commune vient de recevoir une demande préalable de travaux portant sur la toiture et les fenêtres, travaux qui peuvent être subventionnés par l'État.

Quand allez-vous faire confiance aux maires en matière d'urbanisme et leur redonner la capacité d'agir sur leur territoire ? La parole

également essentielle pour notre économie, l'emploi et la survie de nombreuses entreprises. Elle l'est enfin pour réussir la transition énergétique. Construire mieux, c'est bien sûr construire plus durable, plus réversible, plus biosourcé- tous ces nouveaux mots qui sont à la mode, mais qui ont un sens pour le « vivre

Les réglementations s'empilent : chaque époque apporte ses priorités et ses nouveautés. Il est plus que nécessaire de rouvrir le chantier de la simplification du droit de l'urbanisme, et ce au-delà de la dématérialisation, mettre à plat l'ensemble du dispositif, étape par étape, comme l'a proposé l'année dernière la commission des affaires économiques dans le rapport de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Annie Guillemot.

comme nous l'avons fait pour les jeux Olympiques ou Notre-Dame de Paris. La construction et le logement ont besoin de cette « loi olympique » pour sortir de la crise. Il est vraiment dommage que parmi les multiples ordonnances prises ou voulues par le Gouvernement, ce besoin de simplification n'ait pas été retenu. Mais il n'est pas trop tard, madame la ministre

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'espérance que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste porte ce débat sur le devenir de l'éducation prioritaire, l'une des rares politiques nationales visant à lutter contre les inégalités sociales.

70 % des élèves socialement défavorisés ne sont pas scolarisés en REP (réseaux d'éducation prioritaire) ou en REP+. Il est indispensable d'améliorer le dispositif, afin de consolider ces deux objectifs que sont la justice sociale et l'élévation du niveau de connaissances des élèves, en travaillant en réseau, car c'est aussi cela l'intérêt de l'éducation prioritaire. Celle-ci ne se résume pas, même si c'est évidemment très important, à des moyens supplémentaires : elle fait travailler ensemble différents acteurs territoriaux au service de la réussite éducative. Le premier article du code de l'éducation précise clairement que le service public de l'éducation « contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements J'interromps la citation en observant que la réalité est malheureusement tout autre, puisque la France reste en queue de peloton en termes de résorption des inégalités scolaires et sociales.

Le maillage territorial des zones d'éducation prioritaire (ZEP) est aujourd'hui insuffisant. Ce constat est assez largement partagé sur l'ensemble de nos travées : la détermination du label par le collège de secteur n'est pas, ou n'est plus, efficace. Les écoles rurales, qui connaissent elles aussi des difficultés, s'en trouvent exclues. Or il n'y a aucune raison d'opposer les écoles des quartiers et les écoles des campagnes, en prenant des moyens aux unes pour les donner aux autres. Comme le relevait le rapport Mathiot-Azéma, l'éducation prioritaire a fait l'objet d'un recentrage sur les zones de concentration de la difficulté sociale et scolaire, qui met de côté d'autres zones aux problématiques spécifiques, comme c'est le cas de certaines zones rurales l'éloignement des établissements est important, problème qui s'ajoute à d'autres freins existants. Par ailleurs, même en ville, de nombreuses écoles ayant toutes les caractéristiques pour être en REP s'en trouvent exclues, car leur collège de secteur n'en remplit pas les critères. Ainsi, que ce soit à la ville ou à la campagne, ces écoles dites « orphelines » n'ont tout simplement pas accès aux moyens supplémentaires auxquels elles pourraient pourtant légitimement prétendre. Vous annoncez vouloir répondre à ces défis en expérimentant un nouveau dispositif dans trois académies à la rentrée prochaine.

À la rentrée 2021, les trois académies de Lille, Aix-Marseille et Nantes appliqueront la réforme à titre expérimental, et ce jusqu'en 2024, avec un premier bilan tiré en 2023. Qu'arrivera-t-il en 2022 au moment du renouvellement de la carte des REP ? Sera-t-il à nouveau ajourné ? Je rappelle que la révision de cette carte aurait dû avoir lieu en 2019 et qu'elle a déjà été reportée. Nous pensons au contraire que ce zonage devrait être réexaminé maintenant, pour prendre en compte les difficultés engendrées par le confinement du printemps dernier dernier et les dégâts sociaux qu'entraîne la crise sanitaire. La contractualisation qui serait désormais la règle, en lieu et place du travail en réseau, nous interpelle aussi. Nous sommes favorables à une allocation des moyens tenant compte de la réalité concrète mais, d'une part, l'application des différents par les services de l'éducation nationale est souvent très technocratique et, d'autre part, que se passera-t-il lorsqu'au bout des trois années requises les contrats locaux d'accompagnement ne seront pas reconduits ? Les établissements ayant signé un contrat avec le rectorat perdront-ils tous leurs accompagnements spécifiques ? par exemple des dédoublements ? Maintiendra-t-on le dédoublement dans une école qui n'est pas retenue pour mettre en oeuvre un contrat local d'accompagnement (CLA) ? Poser la question revient, malheureusement, à y répondre. Et pourquoi cette durée, pourquoi cette durée, d'ailleurs ? Pensez-vous vraiment qu'il s'agit d'une durée suffisante pour que les différents acteurs parviennent à engager des dynamiques positives ? Beaucoup d'entre nous, ici, vous ont au contraire alertée sur la nécessité d'une stabilisation des équipes pédagogiques, afin de leur donner le temps

une commune rurale de mon département de Seine-Maritime s'est vu refuser l'obtention du label « école du numérique » au motif à peine voilé qu'elle est à classe unique, alors que l'heure est aux regroupements, parfois forcés. D'autres communes qui envisageaient un projet de regroupement pédagogique, avec le maintien de classes dans chacune des communes rurales, ont elles aussi été confrontées au rejet de leur projet par les services académiques, pour lesquels le regroupement ne peut se concevoir que dans un seul lieu, excluant toutes les autres communes, avec les conséquences que l'on connaît. Comment éviter cette forme de pression et s'assurer que l'attribution des contrats ne répondra pas seulement aux exigences académiques, mais aussi à celles des autres acteurs éducatifs de terrain ? Comment élargir les dispositifs permettant de donner plus à ceux qui ont moins ? Voilà la seule question qui devrait se poser, tout particulièrement dans le contexte que nous vivons. Cela passe par des moyens supplémentaires. J'évoquais précédemment la carte scolaire.

aux heures supplémentaires prévues pour soi-disant compenser la baisse du nombre de postes, elles ne sont pas effectuées pour un très grand nombre d'entre elles. Près de 12,5 millions d'euros de crédits dédiés à ces heures supplémentaires n'ont ainsi pas été consommés en 2019.

Moins de 3 % des 2 milliards d'euros consacrés à la formation des enseignants sont destinés à ceux qui exercent en ZEP ; c'est inversement proportionnel aux besoins. De même, il n'est pas du tout pertinent à nos yeux de fondre la prime REP dans la prime d'activité, sauf à vouloir peu à peu utiliser l'une pour pallier l'autre. Il est urgent, à notre sens, de relancer le processus de l'éducation prioritaire. En ce sens, nous proposons de cibler plus finement les établissements, en s'attachant plus fortement au lieu au lieu de vie et en s'appuyant, notamment, sur les données sociales de l'Insee et des services communaux. En intégrant automatiquement dans les REP les écoles situées dans des quartiers prioritaires de la politique de ville ou des communes percevant la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale, en dotant mieux ces écoles, nous éviterions sans doute plus efficacement les dérogations à la carte scolaire. Dans la même perspective, il faut renforcer la formation des enseignants en REP et y affecter plus de remplaçants. Je l'ai dit, cela demande à la fois des moyens de formation et des effectifs en hausse. Dans ce sens toujours, pourquoi ne pas envisager une pluriannualisation des attributions et des retraits de postes ? Voilà qui permettrait par exemple de remédier aux effets de seuil souvent évoqués. Cela inscrirait les équipes pédagogiques dans la durée et permettrait d'anticiper d'éventuels mouvements de population et d'en finir avec ces décisions couperets, qui déstabilisent toute la communauté éducative. aussi, d'accorder des bonifications aux professeurs et de prévoir davantage d'infirmières. Les collectivités locales doivent pouvoir être associées à une réflexion sur l'ensemble de ces sujets.

Deuxième avancée, bien connue : le dédoublement de classes en REP. Désormais, 300 000 élèves de CP et de CE1 sont concernés.

en mathématiques et en français, parce qu'il faut renforcer les compétences pédagogiques de nos professeurs dans ces matières. Certes, les résultats de la lutte contre les inégalités scolaires ne sont pas à la hauteur, et cela d'un double point

passe, bien sûr, par le dialogue social, par la prise en compte des propositions des uns et des autres, donc par la concertation. Différenciation, concertation, sur-mesure : tel

Conformément aux préconisations du rapport Mathiot-Azéma, remis au ministre en 2019, il s'agit de diminuer les effets de seuil induits par la carte de l'éducation prioritaire, jugée trop dichotomique. Des « contrats locaux d'accompagnement » de trois ans, passés entre les rectorats et les établissements, doivent être expérimentés à la prochaine rentrée de septembre dans trois académies. À terme, dès la rentrée de 2022, ces contrats pourraient remplacer l'actuel dispositif des réseaux d'éducation prioritaire, qui concerne plus de 700 collèges et leurs écoles de secteur. Ces contrats devront apporter souplesse et efficacité à l'action des rectorats, qui pourront non seulement sélectionner les établissements susceptibles d'être les plus soutenus, mais aussi distribuer des moyens différenciés selon les besoins locaux : dotation en heures supplémentaires pour organiser de demi-groupes, primes d'attractivité pour les enseignants, décharges destinées à la coordination en équipe, etc. Il s'agit d'une avancée majeure, qui permettra de rompre avec le pilotage national de l'éducation prioritaire. En effet, selon le rapport Mathiot-Azéma, quelque 70 % des enfants défavorisés sont scolarisés dans des établissements qui ne relèvent pas de l'éducation prioritaire. À l'inverse, 25 % des enfants de REP ne devraient pas y être au regard de leur indice de position sociale. Les REP recouvrent des réalités très différentes, selon qu'on se situe dans des régions en fort décrochage économique ou non, périurbaines ou de centre-ville. Ainsi, des écoles, collèges et lycées qui ne bénéficient pas des avantages de l'éducation prioritaire pourront signer ces contrats de trois ans avec clause de rendez-vous.

réforme. Enfin, les écoles dites « orphelines », qui devraient être en REP en raison du profil de leurs élèves, mais qui dépendent d'un collège qui ne l'est pas, pourront également tirer profit du nouveau système. Les critères d'attribution, déterminés à partir d'indicateurs sociaux, ne vont pas changer : le profil du collège et de ses élèves, le nombre de boursiers et les résultats aux évaluations, la proportion d'enseignants titulaires et leur âge moyen entreront toujours en ligne de compte. À cela s'ajoutent de nouveaux leviers, comme le climat scolaire, le taux de décrocheurs, la proximité d'équipements culturels et sportifs. De même, le taux d'attractivité des établissements et le taux de postes partagés seront pris en compte, afin d'intégrer le turnover d'enseignants, néfaste pour la vie d'équipe dans des établissements où la stabilité est primordiale. Pour autant, toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées. Madame la secrétaire d'État, vous nous assurez que la réforme ne va pas être financée sur les crédits dévolus aux REP et aux REP+ et qu'elle sera assurée par des moyens spécifiques. Où comptez-vous trouver ces crédits supplémentaires ? Aux dépens de quels programmes budgétaires ? Enfin, je ne puis que vous encourager à conduire à son terme la réforme annoncée des bourses scolaires, dont une revalorisation se révèle plus que nécessaire au regard de la situation alarmante de notre jeunesse.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l'évoquait ma collègue Céline Brulin, la réforme à venir de l'éducation prioritaire pose de nombreuses questions. Disons-le, nous doutons fortement de la pertinence des réponses que le Gouvernement souhaite apporter aux dysfonctionnements de l'éducation prioritaire. Toutefois, et ce sera ma première remarque, il est difficile pour nous d'avoir un oeil complet sur une réforme dont l'expérimentation commence dans quelques mois et pour laquelle nous avons, finalement, peu d'informations. Mon département, les Bouches-du-Rhône, abrite une des académies tests. Pourtant, nous n'avons encore qu'un regard très flou sur le devenir des 328 écoles maternelles et primaires, ainsi que des 47 collèges aujourd'hui en REP ou en REP+. que nous avons, dans mon département, sur les groupes de travail préfigurant les contrats locaux d'accompagnement sont inquiétants. Ainsi, sur les 72 écoles initialement ciblées dans les Bouches-du-Rhône, seules 39 devraient être concernées. des autres ? Et pourquoi ces écoles précisément ? À ces deux questions, les organisations syndicales n'ont pas obtenu de réponse de la part du rectorat, à l'heure où je vous parle. Ces écoles sélectionnées devraient bénéficier de dix postes et de trente indemnités pour missions particulières. Comment seront répartis ces moyens ? Pour reprendre les termes de Marc Douaire, le président de l'Observatoire des zones prioritaires, « passer d'une logique de politique territorialisée à une politique d'établissement constitue une rupture profonde ». La notion de réseau mobilisant la communauté éducative, le monde associatif et les collectivités territoriales permet de créer un environnement stable et stimulant. Or c'est bien cet aspect social qui est retiré de l'éducation prioritaire. prioritaire. Par ailleurs, c'est une véritable mise en concurrence des établissements qui va être mise en oeuvre. Et comme dans toute mise en concurrence, les perdants sont souvent identifiables en amont de la procédure. On risque donc de se retrouver avec des établissements déjà en difficulté perdant leur label et les moyens qui vont avec. D'ailleurs, madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous éclairer sur les méthodes de quantification et de qualification des projets ? Vous nous aviez présenté certains éléments regroupant des critères sociaux, mais aussi des critères environnementaux comme le taux d'enseignants titulaires, le climat scolaire ou l'indice d'éloignement, mais cela ne répond pas

À quel moment le rectorat considérera-t-il qu'un projet est prometteur ? À quel moment considérera-t-il qu'il a réussi ? Prendra-t-il en compte les « aides extérieures » sur lesquelles certains établissements pourront compter, notamment par le biais d'un surplus d'engagements des collectivités territoriales ? Ne risque-t-on pas, comme le relève Jean-Yves Rochex, de retomber dans des formes de clientélisme comme nous avons pu en connaître sur d'autres sujets ? Pouvons-nous espérer, par exemple, une réforme de l'affectation des enseignants évitant la concentration des jeunes dans des établissements parfois très difficiles ? Autre point sensible : la probable ouverture des dispositifs d'éducation prioritaire aux établissements privés, notamment confessionnels. Après la scolarisation obligatoire à trois ans, ce serait un nouveau cadeau du service public d'éducation nationale au secteur privé. Pourtant, malgré les déclarations rassurantes du secrétaire général de l'enseignement catholique, on ne peut pas dire que l'enseignement privé soit un champion de la mixité sociale ... Le risque que l'on voit venir, c'est que des établissements échangent des exonérations de frais pour les familles tout en se « remboursant » avec la manne de l'éducation prioritaire, la contractualisation avec les rectorats.

On voit bien que, même si l'on pouvait opérer une bascule magique, le 1,4 milliard d'euros aujourd'hui déployé ne suffirait pas à assurer un régime efficace. Or, là, vous proposez d'élargir encore le spectre, quitte à faire bénéficier des établissements qui n'en ont pas besoin. Par ailleurs, on aimerait plus de clarté de votre part. Devant notre commission, vous déclariez ceci : « Quant aux moyens supplémentaires, à ce stade de l'expérimentation, nous allons fonctionner à moyens constants. » Devant nos collègues députés, vous commencez par évoquer « une voie parallèle avec des moyens propres », tout en maintenant le cap des moyens constants. Il est donc bien prévu d'aller chercher les fonds attribués à certaines écoles publiques aujourd'hui pour financer le secteur privé, ainsi que des écoles rurales isolées, qui, s'il est vrai qu'elles ont besoin de de financements dédiés, ne peuvent être rhabillées en déshabillant des écoles urbaines en difficulté. Je conclurai en rappelant un unique chiffre : l'an dernier, sur les 15 postes supprimés dans les Bouches-du-Rhône dans le secondaire, 10 concernaient des sections d'enseignement

est sans appel : 70 % des élèves socialement défavorisés ne sont pas scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, tandis que la Cour des comptes dresse un bilan plutôt décevant de ces politiques. La politique d'éducation prioritaire fait l'objet de nombreuses critiques : notamment un cadre trop rigide ou des effets de seuil qui rendent toute modification de la carte scolaire très difficile. Dès lors, une refonte globale semble nécessaire. En 2019, nos collègues Laurent Lafon et Jean-Yves Roux avaient réalisé un travail de fond, que je salue, sur cette problématique de l'éducation prioritaire, avec la mission d'information sur les nouveaux territoires de l'éducation. Ils constataient qu'un grand nombre d'élèves, pourtant défavorisés, étaient exclus des dispositifs de REP, et plaidaient alors pour une politique de l'éducation prioritaire définie aux niveaux académique et départemental, avec des critères territoriaux, en concertation avec les élus. Cette recommandation trouve son application avec le dispositif des contrats locaux d'accompagnement, qui seront le socle de votre expérimentation, madame la secrétaire d'État. Ce dispositif, qui se veut plus adaptable aux situations locales, permettra de répondre aux écueils des politiques actuelles, en ciblant deux catégories d'établissements : d'une part, des établissements à la lisière des réseaux d'éducation prioritaire ; d'autre part, des établissements ruraux isolés et ne relevant pas des politiques de la ville, dont les besoins sont spécifiques. Cette expérimentation pourrait être une première réponse à la problématique des écoles dites « orphelines », soit 500 établissements. Ils cumulent toutes les caractéristiques des REP, c'est-à-dire un nombre élevé d'élèves boursiers, des parents issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées et un taux de redoublement important. Ces établissements ne peuvent intégrer ces réseaux d'éducation prioritaire, car leur collège de rattachement recrute une population mixte. Ce sont donc quelque 51 000 élèves qui ne peuvent bénéficier des compensations propres à l'éducation prioritaire, par exemple le dédoublement des classes de CP et de Ce dispositif est pourtant efficace pour des élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ces établissements sont tout à fait identifiés par les élus locaux. En intégrant une dimension territoriale à son élaboration, cette expérimentation permettra également de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des écoles situées en zones rurales, grandes absentes des statistiques. Certains territoires, particulièrement en zone isolée ou subissant une crise industrielle ou postindustrielle, voient se cumuler des difficultés sociales qui peuvent avoir des effets scolaires. Et ces dernières ont été aggravées par la crise sanitaire que nous traversons. Dès lors, comment comprendre les fermetures de classes annoncées dans ces territoires, notamment pour les communes de moins de 5 000 habitants ? Ce sont justement ces territoires qui doivent bénéficier d'une attention particulière.

des difficultés sociales et d'apprentissage. Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, si l'idée est de rebattre les cartes pour coller au mieux aux besoins réels des établissements, nous soutiendrons votre expérimentation. Celle-ci ne pourra atteindre ses objectifs qu'en concertation avec les acteurs locaux, et avec des moyens humains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'éducation prioritaire est au coeur de notre promesse républicaine ; c'est l'un des piliers de notre politique en faveur de l'égalité des chances. Le Sénat examinera bientôt le projet de loi confortant le respect des principes de la République : il est bon de se rappeler que c'est d'abord par de tels outils que nous pouvons lutter efficacement contre les séparatismes. Cela ne signifie pas que l'éducation prioritaire doit être pensée de façon figée. Le quinquennat précédent a permis une révision ambitieuse, la première depuis les lois Savary. Élaborée en lien étroit avec les acteurs de l'éducation prioritaire, elle a créé un indice social juste et objectif, élaboré une nouvelle carte de l'éducation prioritaire et impulsé une dynamique reposant sur un travail pédagogique en réseau. Je remercie le groupe CRCE d'avoir proposé ce débat. J'espère que, à son issue, nous aurons des pistes pour répondre aux défis de l'éducation prioritaire : la nécessité d'une meilleure articulation avec la politique de la ville, la défense de la mixité sociale et scolaire, la problématique des établissements dits « orphelins », la revalorisation des personnels à la hauteur de leur investissement, et, bien sûr, la question des établissements ruraux. Il est positif que ce débat fasse une place à leurs spécificités, d'autant plus que, dans certains départements, la carte scolaire de 2021 se constitue dans la douleur, par manque de moyens, ce qui met directement en concurrence des écoles en REP avec des écoles rurales. Dans la Drôme, la rentrée se fera à moyens constants. Pour dédoubler des classes en REP, il faut prendre les postes quelque part. Et souvent, c'est dans les territoires ruraux ! Cette mesure de dédoublement est une bonne chose, mais les moyens pour la mettre en oeuvre n'ont pas suivi. J'espère sincèrement que ce sera l'occasion d'une prise de conscience. Les classes en REP et les classes rurales ont en commun d'avoir des besoins spécifiques, mais ceux-ci ne sont pas les mêmes et ne doivent pas être opposés. Il faut prendre les deux en compte et, surtout, les financer comme il se doit. Nous faisons nôtre également une partie des constats mis en avant pour justifier cette réforme, mais cette expérimentation en vue de transformer l'éducation prioritaire semble créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le premier point qui pose question, c'est sa temporalité très courte. Comment se prononcer sur la pertinence d'une généralisation à partir d'une expérimentation d'un an seulement, alors que les contrats locaux d'accompagnement sont prévus pour une durée de trois ans ? Pourquoi lancer une opération dans la précipitation, alors que nous approchons de la fin du quinquennat ? Cette évolution majeure du système d'éducation prioritaire doit au contraire être pensée dans le temps long, dans une optique de concertation avec les syndicats et la représentation nationale. Les réactions suscitées par l'annonce de cette réforme montrent combien c'est nécessaire. Nous nous interrogeons aussi sur son financement. Madame la secrétaire d'État, vous avez annoncé un budget spécifique de 3,2 millions d'euros dans le cadre de l'expérimentation, dont la répartition dépendrait des contrats signés par les académies. Comment appréciera-t-on si son montant est adapté aux besoins réels ? Quels seront les critères de répartition ? Et sur quel budget cette somme sera-t-elle prise ? Le risque vient également des nouveaux indicateurs de choix des établissements retenus : en plus des critères nationaux, vous avez indiqué que des indicateurs spécifiques « aux mains des académies » seront définis, par exemple le climat scolaire. La conséquence en une dilution des critères sociaux, pourtant au fondement même de l'éducation prioritaire. Cette réforme s'appuie sur une vision de l'enseignement prioritaire contractualisé, émancipé de tout pilotage national au profit d'arbitrages locaux. tel changement conduira fatalement à une rupture d'égalité entre les territoires et à une mise en concurrence des établissements. Nous partageons un constat acteurs et actrices de terrain doivent être mieux associés pour constituer la carte de l'éducation prioritaire. Mais cela n'implique pas la disparition d'un cadre national. du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je vous propose de retourner le problème : au lieu de s'appuyer sur des contractualisations locales, demandons dans un premier temps aux académies quels sont les besoins réels sur le terrain, pour ensuite, à partir de ces remontées, dessiner la carte nationale de l'éducation prioritaire.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie le groupe CRCE d'avoir proposé ce débat. « Le français, la morale, le calcul ! », proclamait Jules Ferry. Sa devise illustrait alors la priorité de l'école élémentaire obligatoire et gratuite l'égal accès de tous aux apprentissages fondamentaux et aux capacités citoyennes. Puis, progressivement, l'école a suivi le cours de l'évolution de la société, marquée par le besoin de spécialisation et de qualification. L'école capable d'offrir à tous l'égalité des chances par le travail, par la motivation par le mérite est venue charpenter l'image de l'école vectrice de l'ascenseur social. La promesse scolaire était alors non plus celle de l'instruction élémentaire pour tous, mais plutôt celle de l'égalité des chances, par le mérite tout d'abord, puis de plus en plus par la différenciation et l'adaptabilité. Ainsi est née en 1981 l'éducation prioritaire, chargée de corriger les maux de la société pour mieux parvenir à l'égalité des chances. Pourtant, quarante ans après sa création, force est de constater que l'éducation prioritaire n'a atteint ni son objectif de mixité ni, surtout, celui de limiter à 10 % les écarts de niveau entre les élèves des zones prioritaires et les autres. Au contraire, plus les élèves empruntent les voies du succès et de la réussite et plus la société leur accorde une offre scolaire de qualité et coûteuse.

Je crois en fait très profondément que l'éducation prioritaire a souffert du non-respect de son principe initial, c'est-à-dire son caractère temporaire. Prévue à l'origine pour quatre ans, sa pérennisation par le zonage a marqué au fer les établissements désignés, accélérant le départ des familles les plus favorisées et le turnover des enseignants. Mes chers collègues, soyons clairs : cette politique était indispensable ; pour autant, nous nous devons de discuter aujourd'hui de la modestie de ses résultats, d'en trouver les causes et de proposer des solutions concrètes. Pour cela, je vous livre aujourd'hui les constats que j'ai dressés. La réduction des effectifs des classes a été et demeure un moyen trop peu souvent utilisé. Les enseignants affectés sont les moins expérimentés, l'absentéisme y est le plus marqué et les contractuels le plus nombreux. De fait, les mesures d'amélioration de l'attractivité de postes et de stabilisation des équipes éducatives ont été atténuées par la rigidité de gestion des enseignants. Il est également nécessaire de souligner l'absence d'autonomie des établissements et de marges de manoeuvre pour les chefs d'établissement. Enfin, la labellisation des établissements en réseau d'éducation prioritaire et l'octroi des dérogations à la carte scolaire ont encouragé les stratégies d'évitement des familles et ont contribué à réduire encore la mixité sociale. Madame la secrétaire d'État, si votre souhait est d'ouvrir le chantier de l'éducation prioritaire, lancez-vous dans la refonte d'un dispositif vacillant et dépassé, en vous détournant d'une politique centralisée à laquelle on vient, pourtant, de vous inviter encore. Ne vous limitez pas à une simple réforme paramétrique du dispositif, faisant fi des erreurs passées. Pour faire réussir l'éducation prioritaire, il vous faudra adapter les modalités de gestion et d'affectation des professeurs afin d'attirer, de stabiliser, de former et de soutenir les équipes. Cette ambition renouvelée impliquera nécessairement une augmentation des postes à profil, le renforcement de la formation, l'affectation d'enseignants chevronnés, des conditions de rémunération plus attractives et des modalités d'affectation spécifiques. Il faudra entrer dans une école du contrat, contrairement à ce qui vous a été dit il y a un instant, avec des contrats de mission destinés à permettre aux professeurs chevronnés de venir servir dans ces territoires difficiles. Pour faire réussir l'éducation prioritaire, il vous faudra aussi adapter l'école à la diversité des territoires et, pour cela, consulter les élus et les équipes éducatives, en les interrogeant sur leur réalité, leur spécificité, en échangeant avec eux sur leurs attentes, leurs difficultés et leurs réussites, les invitant à partager leurs idées, leurs propositions et même leurs revendications. Bref, pour réussir, il vous faut faire du sur-mesure, au plus près des établissements, en laissant la main aux acteurs de terrain. Il vous faut desserrer l'étau de la centralisation et du zonage descendant auxquels on vous a encore appelée, pour permettre aux équipes de terrain de prendre une part active aux esquisses de l'école républicaine de demain. Voilà le chantier de l'éducation prioritaire

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'éducation prioritaire était conçue comme un dispositif temporaire de discrimination positive visant à compenser les inégalités sociales en matière scolaire, en renforçant les moyens de l'éducation nationale en direction des élèves des quartiers défavorisés.

En 2017, le réseau de l'éducation prioritaire couvrait 1 000 collèges, dont 356 en REP+, et 7 000 écoles, dont 2 500 en REP+, pour un coût de 1,6 milliard d'euros. Les principaux critères pris en compte sont le taux d'élèves boursiers, le type de quartier, les catégories socioprofessionnelles et, pour les collèges, le nombre d'élèves ayant redoublé au moins une classe. Toutefois, Toutefois, les moyens déployés manquent souvent leur cible, comme le souligne la Cour des comptes dans un rapport d'octobre 2018. Cette politique ne couvre que 30 % des élèves défavorisés, et les effets de bord sont importants de nombreux établissements en difficulté sont écartés du dispositif ; une école placée en plein coeur d'un quartier prioritaire peut ainsi être exclue du réseau si son collège de rattachement n'en fait pas partie.

Le renouvellement de la politique d'éducation prioritaire depuis 2017 et la réforme en cours visent à remédier à ces problèmes. Parmi les récentes réformes figure le dédoublement des classes de CP, de CE1 et de grande section de maternelle. Le Gouvernement a fait ce choix plutôt que celui du dispositif « Maître+ », plus flexible, visant à renforcer ponctuellement l'encadrement de la classe grâce à un enseignant supplémentaire ou un assistant. Pourtant, les deux dispositifs semblent complémentaires. Des assistants pourraient être déployés dans certaines classes en difficulté pour seconder l'enseignant et améliorer l'accompagnement des élèves. La revalorisation des salaires des enseignants et le renforcement des effectifs du personnel non enseignant sont également des facteurs indispensables au succès du dispositif. La mise en place des classes coopératives donne de bons résultats pour favoriser l'apprentissage du vivre-ensemble et traiter les problèmes de vie scolaire. De même, le dispositif Devoirs faits, déployé depuis 2017 dans les collèges du réseau, est très demandé.

cette expérimentation permettra à certaines écoles, certains collèges et lycées, hors réseaux, de bénéficier au cas par cas de moyens supplémentaires, pour améliorer l'accompagnement des élèves. Certains établissements implantés en milieu rural pourront bénéficier de ce dispositif. Si ses résultats se révèlent prometteurs, sa généralisation permettra aux 500 écoles dites « orphelines », présentant tous les critères d'une école de REP, mais rattachées à un collège hors réseau, d'en bénéficier également. Nous considérons qu'une réforme globale du fonctionnement de l'éducation prioritaire est souhaitable, pour ne pas dire indispensable, au regard de l'insuffisance des résultats du dispositif actuel. Nous devons aller vers un maillage plus souple et plus réactif des écoles et des collèges du réseau ainsi que vers une dissociation des écoles et des collèges.

En conclusion de son ouvrage, le commandant Antoine de Saint-Exupéry s'interroge sur l'avenir du jeune enfant né dans la misère qu'il voit face à lui, dans un wagon de troisième classe en partance pour la Russie Ce qui me tourmente [ ...], c'est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. » L'essentiel est de concentrer nos efforts dès le plus jeune âge, afin d'offrir à chaque enfant, quelle que soit son origine, l'accès à la lecture, à l'écriture et à une maîtrise suffisante du français.

La France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre la condition sociale de l'élève et sa performance scolaire est le plus fort. En d'autres termes, notre système éducatif est l'un de ceux qui reproduisent le plus les inégalités sociales ; et voilà plus de dix ans que notre pays trône dans les hauteurs de ce classement.

Le 25 janvier dernier, et durant les dix-sept jours suivants, deux enseignants du collège Lucie-Aubrac de Givors, au sud de Lyon, ont entrepris une grève de la faim pour demander le classement de leur établissement en REP

Doter en moyens humains et financiers les établissements selon des critères sociaux, alléger les classes pour assurer un meilleur suivi des élèves, renforcer la formation des enseignants : tous ces outils sont cruciaux. Pourtant, les écarts dans la maîtrise des compétences de base en français en troisième sont actuellement de l'ordre de 35 % entre collèges des réseaux Écoles, collèges et lycées pour

exit la logique de réseau entre établissements- désormais, la contractualisation sera de mise, avec des moyens en fonction des besoins des établissements, mais selon des critères établis au niveau national. L'ensemble de ces mesures doit être expérimenté dans trois académies à compter de la rentrée prochaine, en vue d'une généralisation en 2022.

Outre l'évidente contradiction entre ces deux affirmations, la question financière est au coeur du problème. En effet, si la logique de contractualisation est poussée à son terme, avec la volonté d'inclure de nouveaux établissements, le tout sans augmentation significative des moyens,

Ce qui favorise la réussite d'une communauté éducative, c'est normalement la mixité entre des élèves bons et moins bons, issus de milieux plus ou moins aisés. Or le privé assèche certains territoires en attirant dans ses établissements les bons élèves qui peuvent se le permettre. Son action va à l'encontre des principes mêmes d'une politique éducative soucieuse de réduire les inégalités. Dès lors, comment concevoir que ces établissements prétendent à des moyens et des fonds normalement dévolus à des structures en difficulté ? Cette décision est extrêmement problématique. Madame la secrétaire nous ne réduirons pas les inégalités éducatives, qui sont, je le rappelle, les inégalités de revenu, de salaire et de logement, à périmètre financier constant, avec plus de bénéficiaires et en faisant des cadeaux à Il nous faut, à l'échelle nationale, une grille claire et transparente de répartition des crédits, progressive, sur la base de critères socio-éducatifs et de mixité. Pour réduire réellement les inégalités, il faudra transférer des fonds depuis les établissements qui réussissent le plus et qui ont le plus de moyens vers ceux qui sont en difficulté.

La perte du label pour un établissement ou sa fermeture peut faire perdre le statut prioritaire des élèves qui le composaient : c'est absurde ! Qu'importe la structure, ce sont bien les élèves qui ne doivent jamais être perdus de vue ; le véritable enjeu, c'est l'accompagnement individualisé.

et qu'il serait possible d'étendre l'expérimentation à d'autres académies au-delà de ce délai. Cette voie de l'extension est indispensable, car, si l'expérimentation est prometteuse, il est pertinent de l'adapter à d'autres territoires : cette réforme pourrait offrir une plus grande souplesse organisationnelle sur le terrain et un accompagnement plus large que le système actuel. comment articuler ces initiatives et le zonage en vigueur, avec ses seuils REP et REP+ ? Les territoires éducatifs ruraux, les TER, que vous avez mis en place, visent à accompagner globalement l'enfant en mobilisant tous les acteurs en milieu rural, à savoir la communauté éducative et les élus locaux. Cette approche transversale de contractualisation a fait ses preuves pour accompagner l'enfant dans son parcours et renforcer son environnement éducatif. Néanmoins, comment sera-t-il possible d'articuler ces expérimentations avec le maintien du zonage actuel et, ainsi, de faire progresser l'ensemble ?

ont un impérieux besoin de moyens supplémentaires. Je suis favorable au renforcement des moyens dans des territoires pouvant connaître des situations conjoncturelles difficiles, liées à la fermeture d'usines par exemple. Malheureusement, le Pas-de-Calais connaît ces chocs conjoncturels et sociaux ; récemment encore,

Je crains que le renforcement des moyens pour les écoles rurales ne débouche sur le regroupement des établissements et, comme le redoutent les maires, sur des fermetures d'écoles. Il est d'ailleurs à noter que vous avez annoncé votre expérimentation sans concertation préalable avec les élus locaux. Va-t-on assister à des transferts de moyens des ghettos urbains vers les zones rurales, alors que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes ? Les écoles rurales ont besoin de moyens, mais de moyens spécifiques. Les interrogations ont été renforcées par le lancement, en janvier dernier, d'une autre expérimentation : les territoires éducatifs ruraux, au sein des académies d'Amiens, de Nancy-Metz et de Normandie. Ce dispositif entend englober le parcours de l'élève depuis sa petite enfance jusqu'à son insertion professionnelle. Le chevauchement de ces expérimentations augmente l'incertitude pour l'ensemble des acteurs concernés quant à l'approche privilégiée par le Gouvernement pour répondre aux enjeux spécifiques aux écoles rurales. Les contrats locaux d'accompagnement, qui permettent aux recteurs d'octroyer des moyens supplémentaires à certains établissements, suscitent eux aussi des inquiétudes : si l'expérimentation est généralisée, elle signera la fin de la coordination nationale garantissant l'équité dans la répartition des moyens.

Je vous remercie

Si la loi sculpte et garantit les droits, c'est l'école qui peut, patiemment, mais sûrement, façonner, ciseler la clé des chances de surmonter les déterminismes sociaux. Ces chances, ce sont celles de s'épanouir, de s'insérer et de progresser sur l'échiquier de la société. École et République sont donc consubstantielles dans le socle des valeurs qui fondent notre pacte social. Mais elles sont aussi unies historiquement, car c'est la République, la III, au début de la décennie 1880, au Jules Ferry, qui a rendu l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire et l'enseignement public laïc ; et c'est l'école qui, en métamorphosant ses élèves en citoyens instruits et éclairés, a profondément enraciné la République jusqu'à nos jours, si l'on excepte le sinistre épisode de Vichy. Or l'égalité des chances ne se décrète pas ; elle s'élabore pas à pas, mais reste fragile et le fameux âge d'or de la III République doit être nuancé. Après l'école primaire, la poursuite des études y était rare. L'Ancien Régime et les privilèges avaient certes été effacés, mais les castes et les classes perduraient. Mieux valait être bien né pour accéder à des fonctions éminentes. Selon que vous étiez puissant ou misérable, les portes s'ouvraient ou restaient closes. La prolongation de la scolarité obligatoire à seize ans, en 1959, et la création du collège unique, en 1975, avaient aussi pour but l'égalité des droits et des chances. Las, les résultats des élèves sont restés très inégaux et largement liés à l'origine sociale. Est alors née officiellement, en 1981, la politique d'éducation prioritaire. Son principe, la discrimination positive, apparue notamment aux États-Unis dans les années 1960, consiste à donner plus à ceux qui ont moins, à favoriser les défavorisés. Cette politique de différenciation territoriale concerne aujourd'hui un peu plus de 1,7 million d'élèves, soit 20

est-il juste ? Non, malheureusement. Un seul chiffre l'illustre, rappelé de nombreuses reprises : quelque 70 % des enfants socialement défavorisés sont aujourd'hui hors des dispositifs d'éducation prioritaire. La Cour des comptes a d'ailleurs insisté sur cette réalité. Nous connaissons tous, dans nos départements, des écoles ou des collèges avec un public socialement fragile, qui mériterait de bénéficier de moyens supplémentaires.

pour mieux répartir les moyens d'action ? Le système est-il efficace ? Bien des observateurs sont dubitatifs. Les résultats restent modestes, et l'écart demeure malheureusement important, au titre du brevet des collèges par exemple. Le Cnesco pointe à la fois la dilution des moyens et moyens et un mauvais calibrage du zonage des bénéficiaires. Le dédoublement des classes de CP, de CE1 et désormais de grande section, engagé en 2017, peut apporter une réponse appréciable, même s'il est trop tôt pour crier victoire. Certains enseignants insistent d'ailleurs sur le revers de la médaille : certains élèves perdent une relative aptitude à l'autonomie.

également à l'esprit une catégorie d'élèves dont nous n'avons pas parlé : les lycéens des zones rurales dépourvues de lycées, qui partent tôt le matin pour rentrer tard le soir. Peut-on parler d'égalité des chances pour ces jeunes, qui passent deux à trois heures par jour dans les transports ? Non !

la politique d'éducation prioritaire, mise en place dans l'urgence en 1981 pour « donner plus à ceux qui ont le moins », devait faire réussir tous les élèves. C'est sans doute ce défi qui m'a donné envie, cette année-là, de devenir enseignante. Jusqu'à mon élection au Sénat en septembre dernier, j'exerçais ma profession dans un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, un Rased, d'abord à Mulhouse, puis dans le Sundgau, un territoire rural du sud du Haut-Rhin. Lorsque cette structure n'a plus été en mesure de remplir ses missions auprès des élèves, mon rôle a consisté à accompagner les enseignants qui avaient mobilisé et épuisé les moyens mis à leur disposition pour tenter d'aider les élèves dépassés par les attentes de l'école. accompagné des parents en détresse : vers qui se tourner quand le milieu rural se révèle être un désert sanitaire et quand la première antenne de soins médico-psycho-pédagogique se trouve à plus d'une heure de route, avec une liste d'attente de deux années J'ai ainsi vécu sur le terrain l'évolution de cette politique publique, avec laquelle a précisément commencé ma vie professionnelle, et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui vous faire part de mon expérience. Mon premier constat, c'est que jamais, durant ma carrière, l'éducation nationale n'aura pris en compte la ruralité et ses spécificités. La politique de l'éducation prioritaire a été collée sur la politique de la ville, et de larges moyens ont été affectés aux zones urbaines, au détriment des autres territoires. Aujourd'hui, on se retrouve avec une fracture entre l'école des villes et l'école des champs, alors que plus de dix millions de jeunes de moins de 20 ans vivent en zone rurale et que 75 % des élèves socialement défavorisés ne sont pas scolarisés en REP ou en REP+. Depuis les années 1980, l'école en milieu rural fait l'objet d'une politique par défaut. Depuis quarante ans, elle sert de variable d'ajustement de la politique de la ville, qui a concentré un maximum de moyens sans avoir produit les résultats escomptés. À l'arrivée, ceux qui en font les frais sont ceux que l'on croyait épargnés : des élèves qui vivent dans des territoires sans équipements culturels ou socio-éducatifs, scolarisés dans des classes à multiniveaux, soutenus à bout de bras par des enseignants qui n'ont ni la formation adéquate ni la disponibilité nécessaire pour faire face à la grande difficulté scolaire et aux troubles du comportement qui explosent partout depuis une dizaine d'années. Mon second constat est encore plus alarmant. Les professionnels sont à bout de souffle, épuisés, parfois même soupçonnés d'incompétence, alors qu'ils sont simplement dans l'impossibilité d'apporter des réponses adéquates au sein même de l'école,

dans toutes les écoles. Il faut réduire le nombre d'élèves par classe partout et non uniquement dans les zones dites « sensibles ». Il faut renforcer les réseaux de professionnels spécialisés qui interviennent à l'école aux côtés des enseignants. Ces personnels sont à même de traiter des situations de détresse affective et éducative par un suivi personnalisé de chaque élève en difficulté et de sa famille. Madame la secrétaire d'État, il faut prévenir la difficulté scolaire et la traiter à temps aujourd'hui,

à détruire, mais au contraire à renforcer et à élargir les moyens et les dispositifs permettant de mieux accompagner nos élèves, nos familles et nos professeurs.

Je vais maintenant tenter d'aborder l'ensemble de vos questions par un propos général, dans lequel vous trouverez, je l'espère, l'ensemble des réponses que vous attendez. Depuis 2017, Jean-Michel Blanquer a fait beaucoup pour l'éducation prioritaire. Je peux citer, par exemple, le dédoublement des classes de CP et de grande section, aujourd'hui à taux plein, qui concernent 300 000 de nos élèves en éducation prioritaire. Je suis en train, avec le ministre, de dédoubler les classes de grande section. Nous allons progressivement monter en puissance pour atteindre cet objectif dès 2022.

direz peut-être que je répète les propos du Premier ministre, mais je suis très attachée aux territoires et je ne m'arrête pas à la descente des trains dans les grandes villes

pour accompagner tous nos élèves, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle, en mobilisant l'ensemble des forces vives sur nos territoires.

que je porte au secrétariat d'État, à la suite de tout ce qui a été fait par le ministre Jean-Michel Blanquer. Bref, tout va bien ! Revenons maintenant à ce qui a mobilisé bon nombre de vos questions, à savoir les contrats locaux d'accompagnement.

l'éducation prioritaire concerne aussi la ruralité, laquelle a été très mal desservie à l'occasion de ce dernier zonage. C'est donc sur la base de l'ensemble de ces constats que j'ai décidé de lancer cette expérimentation.

nous avons déjà mené une trentaine d'audiences avec l'ensemble des organisations syndicales. J'ai également à coeur de travailler avec tous les élus. J'ai été moi-même une élue municipale, une élue régionale et une parlementaire ne sais que trop combien il est important de travailler en concertation avec l'ensemble des élus. Cette expérimentation a donc été annoncée, travaillée et préparée avec les élus et les organisations syndicales, et nous continuerons à agir le calendrier, l'expérimentation a été annoncée au mois de novembre dernier ; depuis lors, nous avons installé un comité de pilotage.

J'ai très clairement mandaté ces dernières, parce que je souhaite faire entrer de nouveaux publics et de nouveaux territoires dans cette expérimentation. Je leur ai donc demandé d'être particulièrement attentives à nos écoles orphelines, à nos lycées professionnels et à nos territoires ruraux.

je le répète, mais une voie parallèle. Cela signifie que je ne touche pas au zonage existant, c'est-à-dire aux REP et aux REP+, non plus qu'aux moyens qui sont alloués à cette carte. C'est en ce sens que j'ai parlé de moyens constants. Néanmoins, l'expérimentation menée en parallèle bénéficie d'un budget spécifique, de 3,2 millions d'euros.

complètement différent, qui sort du zonage et de la logique du tout ou rien, pour aller vers plus d'équité, de justice, de souplesse et une meilleure allocation des moyens,

récurrente et progressive des effectifs. Nous avons ainsi perdu environ 65 000 élèves. Pour autant, nous n'avons cessé d'augmenter les moyens, en particulier sur le premier degré,

En effet, je travaille activement à restructurer nos fonds sociaux. J'ai constaté que, dans bon nombre de nos établissements, ceux-ci ne sont pas consommés ou sont sous-consommés.

ou des réinscriptions, solliciter les familles, qui, dans le contexte si particulier que nous traversons, sont de plus en plus nombreuses à avoir des besoins et, malheureusement, ne connaissent pas ces dispositifs ou n'osent pas les demander. J'étudie également, avec Olivier Dussopt,

à un nouveau mode de distribution de ces petits-déjeuners dans nos établissements. Je reviens aux contrats locaux d'accompagnement. Vous considérez que leur temporalité est trop courte

avec l'objectif de l'améliorer. C'est le principe de l'expérience et du tâtonnement : on fait, puis on s'améliore. Ces contrats locaux d'accompagnement sont conclus pour trois ans, avec, peut-être, une clause de rendez-vous. « Peut-être » parce que,

Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. » C'est précisément ce à quoi je m'emploie au secrétariat d'État à l'éducation prioritaire pour assurer l'élévation générale du niveau de nos élèves et la réussite de tous nos enfants sur tous nos territoires. Nous en